Avant de passer au vote sur l'ensemble du texte, je vais donner la parole à ceux de nos collègues qui ont été inscrits par les groupes pour expliquer leur vote. J'indique au Sénat que, compte tenu de l'organisation du débat décidée par la conférence des présidents, chacun des groupes dispose de sept minutes pour ces explications de vote, à raison d'un orateur par groupe.

Je l'avais déploré lors de la discussion générale en ouverture de nos débats, le partage des crédits, parfois pour des actions identiques, entre plan de relance et missions budgétaires classiques, crée du trouble et une absence de lisibilité. Cela a pu donner lieu à des votes déstabilisant l'équilibre budgétaire ou la philosophie des missions. À défaut de les cautionner, nous pouvons tous admettre que ces votes ont permis de mettre en exergue des difficultés réelles ou ressenties. Il m'est impossible de revenir sur toutes les modifications apportées au texte Je retiendrai trois grandes lignes, qui constituent en quelque sorte la philosophie sur laquelle nous aurions pu fonder notre plan de relance. Tout d'abord, comme l'ont dénoncé Philippe Dallier, Dominique Estrosi Sassone et Marc-Philippe Daubresse, nous avons travaillé à une politique du logement plus efficiente, en ayant à l'esprit que, « quand le bâtiment va, tout va » : prolongation du PTZ jusqu'en 2024 ; suppression du recentrage du dispositif Pinel sur les seuls logements collectifs ; taux réduit de TVA pour l'ensemble des livraisons d'immeubles réalisés en vue d'un bail réel solidaire.

et, demain, dans la relance par leur capacité d'investissement, nous avons choisi de préserver leurs capacités financières : contemporanéité du FCTVA compensation des pertes de CVAE des départements et des EPCI ; reconduction en 2021 du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales du bloc communal. Enfin, nous avons soutenu un certain nombre de dispositifs visant à conforter les fonds propres des entreprises en mobilisant l'épargne privée ouverture du PEA-PME aux actions des sociétés de capital-risque ; création d'un IFI-PME ; hausse du taux majoré de réduction d'impôt sur le revenu pour la souscription au capital des PME.

forêt et affaires rurales », nos rapporteurs spéciaux n'ont pas réussi à trouver de réponses aux problèmes structurels qu'ils dénoncent et qui se traduisent par une perte de compétitivité. asile et intégration » ne permettront pas à l'État de contrôler l'immigration en amont. Les mesures proposées visent uniquement à la rendre plus acceptable, aussi bien pour les personnes accueillies, à qui nous devons le respect en tant que personnes humaines, que pour celles qui en subissent les nuisances. Le montant des dépenses de l'aide médicale de l'État vient de dépasser le milliard il serait peut-être temps de considérer la proposition que nous avons faite en première partie d'une aide centrée sur un panier de soins et sur la prévention. Le Sénat s'est également opposé, avec force, à la remise en cause de la parole de l'État. Que l'engagement ait été pris à l'égard des collectivités- mécanisme de compensation de la perte des recettes de taxe d'habitation -ou d'acteurs économiques- les exploitants d'installations photovoltaïques de grande taille -, notre position est identique : l'État ne peut pas revenir de manière unilatérale sur ses engagements sans renforcer le contexte de méfiance. Il me semble que nous n'avons pas besoin de cela Au moment de conclure, nous avons bien évidemment le regret qu'un certain nombre de questions posées soient restées sans réponse. Nous déplorons également que le débat démocratique ait souffert de l'absence de certains ministres, qui ne sont pas venus défendre leur budget. Ils n'ont pourtant

C'est d'autant plus regrettable que, lorsque les ministres titulaires sont venus, les échanges ont été très nourris. Je pense ici à la discussion du budget de l'éducation nationale ou de celui de l'agriculture Ces critiques, monsieur le ministre Dussopt, ne vous sont absolument pas adressées. Au contraire, nous avons apprécié la courtoisie et la précision de vos réponses, toujours en bonne intelligence. J'adresserai également des remerciements, doublés de félicitations, à notre rapporteur général, Jean-François Husson.

à la crise économique que nous traversons. Il est également conforme à notre vision de l'écologie : une écologie positive, et non pas punitive, une écologie accessible à tous. Cependant, nous demeurons inquiets quant au niveau de dette qu'il lègue aux générations futures. Nous avons bien compris qu'un comité Théodule trouver une solution à cet argent qui n'est pas magique. C'est un enjeu de société. Il serait opportun d'y associer le Parlement afin d'éviter de renforcer encore un peu plus le sentiment d'un gouvernement d'experts. La parole

Ce sont les conséquences des dépenses que nous avons votées et des recettes qui ont manqué. Le passé, ce sont les stigmates budgétaires du « quoi qu'il en coûte », dont nous avons fait notre mot d'ordre collectif. L'avenir, c'est l'horizon qu'il est de notre devoir de dessiner ensemble pour la France. C'est l'impérieuse nécessité de renouer avec la croissance, notamment en accélérant notre transition écologique. C'est l'innovation scientifique et la réindustrialisation des territoires, l'objectif étant d'adapter notre modèle de développement aux enjeux de demain. En un mot, ce budget est placé sous le signe de la relance. Dans cette période que nous savons si particulière, alors que nous doutons de nos choix de société, dans un monde qui se bipolarise, nous devons être à la hauteur. L'enjeu consiste à bien articuler ces deux temporalités, le passé et l'avenir. D'une part, il s'agit de répondre au besoin de protection exprimé par les Français au cours de la crise sanitaire et économique. La colère sociale monte et fait planer une menace inquiétante sur notre avenir. D'autre part, il s'agit de ne pas laisser croire que l'ambition de notre politique ne se mesure qu'à l'aune des deniers publics débloqués pour la relance. Les efforts collectifs ne se jaugent pas uniquement en argent public. La dette obère l'avenir des jeunes générations, déjà obscurci par l'épidémie. La situation très inquiétante de nos finances publiques en cette fin d'année doit à cet égard nous alerter. Notre taux d'endettement a bondi de 20 points en moins d'un an. Les dépenses publiques représentent près des deux tiers de la richesse nationale. C'est du jamais vu Cela étant, je l'ai dit, on ne peut pas analyser le projet de loi de finances pour 2021 en se contentant de commenter les principaux indicateurs macroéconomiques. L'important est de déterminer si le budget du plan de relance nous met, oui ou non, sur de bons rails pour l'avenir. Pour cela, nous devons reparamétrer notre grille d'analyse. L'exemple de la dette suffit à le prouver : alors que, en 2020, l'État s'est financé par l'emprunt plus que par l'impôt et que la dette n'en finit pas d'enfler, la charge de la dette, elle, continue de baisser. Cette bizarrerie est le résultat du contexte macroéconomique, les taux étant maintenus artificiellement bas par la Banque centrale européenne. Il est facile, même logique, d'y voir une certaine incitation à l'endettement. Or le risque d'une remontée des taux, longtemps agité comme un chiffon rouge, se précise. Dans un article paru il y a un mois dans, l'économiste Pierre Cahuc explique pourquoi le miracle de l'argent gratuit pourrait bientôt cesser, du fait de la remontée des taux d'intérêt réels, interrogeant ainsi notre stratégie d'endettement. Cette hypothèse nous oblige à changer de logiciel : certes, on ne peut pas se satisfaire d'une analyse des indicateurs classiques, mais on ne peut pas non plus continuer à faire comme si l'argent allait demeurer si bon marché, à cause d'une épargne qui tendrait à se réduire dans les années à venir. Mais, pour l'heure, la situation est tout autre. Grâce aux mesures d'urgence et du fait des restrictions sanitaires, les Français ont épargné plus de 90 milliards d'euros supplémentaires cette année.

L'enjeu collectif, me semble-t-il, est donc aujourd'hui de mobiliser utilement cette épargne privée afin de consolider les dépenses publiques. Certes, l'avenir de nos commerces et de nos restaurants dépendra largement de la propension des Français à consommer, comme lors du premier déconfinement.

Il y va de notre capacité à renouer avec la croissance sans recourir ni à l'endettement ni aux hausses d'impôts. Il y va aussi de l'adhésion des Français à la dynamique de la relance, voire de notre cohésion. Le projet de loi de finances pour 2021 prévoit des dispositifs intéressants pour mobiliser cette épargne, je tiens à le saluer. Je pense notamment à la garantie pour l'investissement dans nos PME et nos ETI permettant de renforcer leurs fonds propres et leur capacité d'investissement,

Je pense enfin à la mission « Recherche et enseignement supérieur », dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur avec mon collègue Jean-François Rapin. Les crédits de cette mission donnent une ossature budgétaire à la loi de programmation de la recherche que nous avons récemment adoptée. Ils concrétisent notre engagement en faveur d'une croissance plus durable, en phase avec les enjeux de compétitivité que la France ne saurait ignorer. Le retour à une forme de croissance est une impérieuse nécessité. C'est la seule façon pour nous de retrouver la maîtrise de notre destin national et de réinventer notre souveraineté.

face à une Amérique en surchauffe et une Asie en accélération continue, nous avons besoin d'un État protecteur, en pointe sur le régalien, juste en appui dynamique sur le reste. En conclusion, mes chers collègues, permettez-moi de vous faire part d'une conviction la réussite de la relance dépend moins des crédits que nous voterons que de notre capacité collective à obtenir des résultats tangibles dans les territoires. Il y va de l'adhésion des Français à ce projet. Dans cet élan collectif, la chambre des territoires doit jouer un rôle clé. C'est pourquoi, tout en saluant le travail de M. le rapporteur général, je regrette que le Sénat n'ait pas adopté les crédits de certaines missions pour lesquelles nous devons réarmer l'État. C'est notamment le cas des missions « Immigration, asile et intégration », « Ces crédits sont en effet essentiels pour préparer notre pays aux défis qui l'attendent. Malgré cela, nous voterons le projet de loi de finances pour 2021, tel qu'il a été amendé par le Sénat, en soutien, monsieur le ministre, au plan de relance prévu par le Gouvernement et attendu par nos territoires. La parole

pas parvenus à convaincre de l'impérieuse nécessité de réformer très profondément la politique fiscale mise en oeuvre par le Gouvernement

l'extension de la garantie jeunes à 50 000 jeunes supplémentaires, mais nous savons que cela ne sera pas suffisant. Par ailleurs, nous doutons de la capacité des missions locales, qui sont pourtant à pied d'oeuvre dans nos territoires, à mettre en oeuvre ces garanties nouvellement budgétées.

Malgré les crédits de la politique de la ville, les habitants de ces quartiers bénéficient en effet de bien moins d'argent public que la moyenne. Nous parlons beaucoup des territoires ruraux ici, et nous avons raison,

entendus. Elles sont soit reportées, comme l'instauration d'une redevance sur les engrais chimiques azotés, soit dénaturées, comme le malus pour l'achat d'un véhicule lourd, qui ne concernera finalement que 2 % des véhicules, soit tout simplement rejetées.

Le rapporteur général, qui n'est pas non plus de mon bord, a dit, lui, que l'ambiance était plombée. Il s'est d'ailleurs réjoui, avec l'honnêteté qui le caractérise, que notre débat soit passé sous les radars grâce à l'actualité chargée. C'est dire si nous pouvions en être fiers

est à M. Jean-Claude Requier, pour le groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen. Monsieur le président,

Le volume d'amendements déposés a doublé en trois ans, avec près de 2 800 amendements déposés cette année, preuve que le Sénat s'est voulu force de proposition. C'est donc un texte particulièrement dense sur lequel nous nous apprêtons à voter, non plus par un scrutin solennel à la tribune, comme c'est l'usage, mais par un scrutin public ordinaire, du fait des restrictions sanitaires. Il est vrai que la mission « Plan de relance » aura beaucoup contribué à la multiplication des propositions, brouillant même parfois la clarté et la lisibilité de la discussion budgétaire, du fait de la nature transversale des outils de relance économique portés par le Gouvernement. Mais cette mission est naturellement indispensable pour soutenir notre économie, dans un contexte historiquement dégradé. Bien sûr, la trajectoire budgétaire initialement prévue par le Gouvernement pour le quinquennat n'a plus lieu d'être. Cependant, la baisse progressive des impôts dits « de production » reste la grande mesure fiscale de ce budget. Déjà annoncée avant la pandémie, elle est aujourd'hui devenue l'un des grands axes de la politique économique du Gouvernement, dans le but légitime d'améliorer la compétitivité de nos entreprises. Le Sénat a adopté cette réforme, tout en veillant à en limiter les effets secondaires, en particulier pour les finances des collectivités locales. Les débats techniques

Par ailleurs, sujet désormais récurrent, la contribution exceptionnelle sur les contrats d'assurance adoptée par notre assemblée se comprend comme une mesure de solidarité nationale, alors que l'on a constaté en 2020 une baisse de la sinistralité du fait des mesures de confinement. Le Sénat a également adopté certaines propositions habituelles de sa majorité, comme le relèvement du plafond du quotient familial. En revanche, il a suspendu l'application du jour de carence pour les agents publics dont l'arrêt maladie est directement lié à l'épidémie de covid-19, comme c'est le cas pour les salariés du secteur privé.

Pour sa part, le RDSE se réjouit de l'adoption de certaines de ses propositions, telles que l'exonération d'impôts pour les organismes de foncier solidaire, l'extension de la déduction pour aléas aux sociétés exerçant une activité agricole dite « prépondérante » et du crédit d'impôt famille aux travailleurs indépendants, la facilitation des fusions de sociétés agricoles, la fiscalité incitative sur les biocarburants, la mobilisation de la contribution climat-énergie en faveur des collectivités engagées dans la transition énergétique, la compensation des effets négatifs pour les collectivités de la réforme de la taxe d'habitation, ou encore la préservation des finances des départements et des ressources affectées aux chambres de métiers et de l'artisanat. La mission « Plan de relance », dont le détail ressemble surtout à un ensemble de crédits supplémentaires alloués aux différents ministères par le biais de trois grands programmes de portée générale- « Compétitivité », « Écologie » et « Cohésion » -, aura sans surprise incité à demander que s'ouvrent plus grand les cordons de la bourse.

je salue la suppression quasi unanime de l'article 54 , qui prévoyait la baisse du tarif de rachat de l'électricité d'origine photovoltaïque. Nous espérons que le Gouvernement en tiendra compte dans la navette. Concernant la mission « Relations avec les collectivités territoriales », avec mes collègues Maryse Carrère et Christian Bilhac, nous avons fait adopter l'inclusion des investissements touristiques dans le périmètre de la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL), ainsi qu'un assouplissement des règles de répartition de la dotation de solidarité communautaire. Nous avons également rétabli les anciennes règles, plus équilibrées, de compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements. Sur la politique du logement, nous avons abondé de 50 millions d'euros le programme d'aide à Action Logement et supprimé une disposition potentiellement préjudiciable aux ressources de cet Le PTZ serait quant à lui prorogé jusqu'en 2024. Sur l'initiative de ma collègue Nathalie Delattre, nous avons oeuvré en faveur du soutien à l'enseignement technique agricole, qui peut relever de la double tutelle du ministère de l'agriculture et du ministère de l'éducation nationale.

Aujourd'hui, près de la moitié du budget de l'État est donc financée par l'endettement. La suspension des critères européens est justifiée, dans le contexte exceptionnel que nous connaissons, mais le poids de la dette va nous poursuivre pendant de très longues années.

dans la liberté et la diversité de notre groupe, nous nous partagerons entre trois votes pour et une majorité d'abstentions. La parole est

d'abord, nous ne pourrons pas nous adresser au ministre Le Maire, qui est pourtant chargé de l'économie et de la relance. Il est vrai qu'il en a été de même du ministre Véran pour la loi de financement de la sécurité sociale. D'accord, les gestes barrières sont importants, mais quand même !

Merci, monsieur le ministre Dussopt, pour votre participation et votre comportement politique, même si je regrette la présomption d'avis défavorable sur nos amendements ! Ce budget est davantage celui d'un fidèle serviteur de l'accumulation du capital celui d'un État souverain où le libre développement de chacun est la condition du libre développement de tous. Mes chers collègues, je me permets simplement de vous le rappeler en toute solennité : le bon sens voudrait que nous ne répondions pas à une crise qui accroît drastiquement nos dépenses par d'autres dépenses. Notre groupe n'a eu de cesse de vous proposer de nouvelles ressources fondées sur l'équité fiscale, afin d'entraver l'accroissement des inégalités que la crise sanitaire continue de renforcer. Or, alors que nous avons débuté les débats autour de ce budget il y a maintenant plus d'un mois, nous avons beau chercher, nous ne trouvons pas ! Nous ne trouvons pas vos propositions visant à rétablir l'équité fiscale entre les petites et les grandes entreprises. Nous ne trouvons pas non plus vos mesures garantissant l'égalité entre les commerces de proximité et les géants du commerce en ligne, qui se sont largement enrichis pendant la crise. Nous vous avons bien proposé une meilleure progressivité de l'impôt sur les sociétés, avec à la clé une baisse d'imposition pour les petites entreprises, vous avons proposé une contribution des géants du numérique et un accroissement de la taxe sur les marchés financiers et sur les versements de dividendes, mais vous n'en voulez pas. Aucun nouvel impôt sur la richesse Il n'y a pas d'argent magique, mais, des décisions magiques, il n'y en a pas non plus ! Non, le véritable problème est moins l'argent que sa redistribution ! Trop souvent, vous pensez aux réductions d'impôts. Crédits d'impôt par-ci, crédits d'impôt par-là ! Mais, alors, allez-y, supprimez tous les impôts sur les entreprises, lâchez-vous ! Mais ça ne marchera pas. Tout le monde le sait, mais on continue ! Arrêtons de vouloir installer le pays dans le cercle infernal de la relance par la dette et de la dette pour la relance ! Entre la majorité de l'Assemblée nationale et celle du Sénat, il y a certes des différences, mais il y a un point commun

faits aux grandes entreprises sur le dos des budgets locaux produira des effets de bord renforçant son injustice. Les collectivités ne sont pas traitées à égalité face aux conséquences de la crise ; surtout, elles ne sont pas assez soutenues. Nous avions bien fait des propositions qui auraient permis de réellement les soutenir, au regard des milliards de pertes engendrées par la baisse de leurs recettes et la hausse de leurs dépenses. Mais la majorité a préféré les décortiquer, révélant ainsi des contradictions, voire des antagonismes entre les beaux mots et les actes. Le choix est clair : au levier d'action publique qui a une légitimité démocratique, à l'expérience locale, on préfère les logiques du marché privé, on préfère fabriquer des clients consommateurs plutôt que des usagers citoyens. Le général de Gaulle, qui est souvent cité, nous rappelle ce qu'est un véritable plan : « Il Il embrasse l'ensemble, fixe les objectifs, établit une hiérarchie des urgences et des importances, introduit parmi les responsables et même dans l'esprit public le sens de ce qui est global, ordonné et continu, compense l'inconvénient de la liberté sans en perdre l'avantage. » Eh bien, mes chers collègues, ce n'est pas un plan que vous allez voter ! Où sont les véritables objectifs ? Quelle est la priorité ? 7 milliards d'euros à l'énergie en voie de nouvelle marchandisation, contre 800 millions pour les plus pauvres. Mais c'est se mettre une balle dans le pied que d'acter que le développement durable soit mieux doté que la lutte contre la pauvreté ! Une aide de 150 euros pour les allocataires des minimas sociaux, une fois, sur un mois, ni plus ni moins ! Nous avions pourtant proposé de baisser la TVA sur les biens de première nécessité pour contrer cette pauvreté galopante, mais vous vous êtes cachés derrière la fatalité de l'« harmonisation européenne comme si nous ne faisions pas partie de l'Europe ... Mes chers collègues, ce budget manque cruellement de vision, d'espoir et de créativité. Ce gouvernement promettait un nouveau monde ; nous récoltons finalement les mêmes recettes, inlassablement. L'Institut des politiques publiques confirme d'ailleurs que, dans votre budget, « les entreprises qui ont le plus pâti de la crise ne bénéficieront pas particulièrement du plan de relance ». Pour toutes ces raisons, nous sommes amenés à dire non à ce budget. Une crise sanitaire ? Vite, baissons les impôts des entreprises de 10 milliards Sur les dix prochaines années, 100 milliards d'euros vont échapper à l'État, monsieur le ministre. Ce sont 100 milliards qui vont manquer à la santé, 100 milliards qui vont manquer aux transports en commun, 100 milliards qui vont manquer pour une politique sociale ambitieuse, 100 milliards qui vont manquer pour l'écologie et les projets des collectivités territoriales À croire que notre pays est devenu un régime de faveur, où seuls ceux qui participent au capital productif méritent des droits. Vous refusez de constater que ce plan constitue- je cite encore l'Institut des politiques publiques -une « confiance aveugle dans les politiques structurelles et de l'offre » et qu'il La relance n'existera pas, mes chers collègues, tant que la diminution de l'investissement public, qui s'est effondré de 26 % au premier semestre, ne sera pas compensée. Si les finances des collectivités sont en berne, la relance de la croissance le sera aussi. J'avais abordé, en introduction de l'examen de ce budget, la nécessité d'ouvrir des perspectives, de donner un horizon, du fait de cette situation difficile pour notre économie, mais surtout pour les gens. Pourtant, vous vous entêtez dans une politique de l'offre injuste et inefficace. Les Françaises et les Français, en contrepartie de la dette, à quoi ont-ils droit maintenant ? Ils ont le droit à un chantage aux réformes dites « structurelles » : réforme des retraites, baisse des dépenses et des services publics, réforme de l'assurance chômage. Ce plan ne relance rien ; il signifie une politique sans partage des pouvoirs et des richesses, autoritaire et régressif. Nous sommes convaincus que ce budget n'est pas un budget de crise face à la crise. Il vient une fois de plus déléguer la souveraineté de l'État à la technoscience et au marché. Nous nous y opposons donc. La parole est

par des budgets en constante augmentation que l'on juge les résultats d'une politique. Nous considérons au contraire qu'il faut continuer les efforts pour que, structurellement, nous adaptions nos dépenses aux recettes dont nous pouvons bénéficier. Il n'est pas pensable de continuer indéfiniment à dépenser plus que l'on n'encaisse. Bien entendu, nous ne pouvons faire abstraction du contexte dans lequel nous nous trouvons ni de la nécessité de mettre en oeuvre des actions de relance économique. On voit bien

des effectifs. Il importe de soutenir l'enseignement agricole, facteur d'aménagement du territoire et de dynamique des territoires ruraux. Cela

La France est pourtant un grand pays maritime ; nous devons affirmer cette vocation maritime, ce qui ne pourra se faire que par une politique cohérente. Certes, un ministère de la mer a été institué, mais

mais le Gouvernement a choisi de continuer sa route. Certes, il prend des mesures indispensables, mais sans dévier de sa politique. À l'issue de nos débats, nous ne voterons pas ce budget, car nous avons la conviction que la crise sanitaire, économique et sociale aurait nécessité de profonds changements. Or force est de constater que la majorité sénatoriale a elle-même inscrit ses pas dans ceux du Gouvernement. Manque de soutien aux victimes de la crise, abandon de la jeunesse face à la précarité, absence de volontarisme en matière de transition écologique, fragilisation des collectivités territoriales, refus d'accroître la contribution fiscale des plus riches comme des grandes entreprises et, de ce fait, creusement des déficits : voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous reconnaître dans ce projet de loi de finances, ni avant ni après sa modification par le Sénat. L'examen de la nouvelle mission « Plan de relance » a été particulièrement révélateur. Si plusieurs de nos amendements ont été adoptés, pour les outre-mer, la culture, le logement, la rénovation urbaine et l'aménagement du territoire, c'est bien parce que le plan de relance du Gouvernement s'avère insuffisant et incomplet. Il se contente d'accentuer la politique de l'offre menée depuis trois ans contre vents et marées. D'autant que ce plan de relance a déjà bien rétréci

cette action sur la compétitivité à moyen terme restera inefficace faute d'être mieux ciblée et davantage conditionnée, surtout faute d'être accompagnée d'un soutien beaucoup plus fort à la demande sur le court terme. Il manque un vrai plan d'urgence à ce budget. D'ailleurs, celui-ci n'est-il pas déjà caduc ? Le Gouvernement s'apprête en effet à introduire de nouvelles mesures à l'Assemblée nationale, et nous n'attendrons sans doute pas très longtemps en 2021 pour voir arriver un premier projet de loi de finances rectificative. Aujourd'hui, Gouvernement et majorité sénatoriale se réjouissent de la baisse des impôts de production. Le Premier ministre lui-même a jugé utile de faire une déclaration qui en dit long : « Le Le plan de relance n'est pas un cadeau fait aux entreprises, c'est un cadeau à la France pour relancer l'économie. » Pour notre part, à l'instar de nombreux économistes, nous nous interrogeons sur l'utilité de ces baisses d'impôts pour les entreprises, sur leur pertinence, leur efficacité, leur coût pour les finances publiques et leurs conséquences pour nos collectivités locales. Ces baisses d'impôts profiteront-elles particulièrement aux entreprises qui ont subi le choc le plus important du fait de la crise sanitaire ? Permettront-elles la réindustrialisation de notre pays ? Sont-elles vraiment l'outil de relance le plus adapté après la crise que nous connaissons ? Permettez-nous d'en douter. Quant au refus obstiné du Gouvernement de faire contribuer fiscalement les plus fortunés, dont chacun reconnaît que l'épargne s'est pourtant considérablement accrue, il a lui aussi trouvé un écho favorable et assez prévisible auprès de la majorité sénatoriale. D'ailleurs, comme Julien Bargeton le rappelait, vous avez voté ensemble en faveur de la première partie de ce projet de loi de finances. Pourtant, toutes les études montrent que la crise a exacerbé les inégalités. Ce sont les Français les plus modestes qui sont les plus durement touchés par la dégradation de la situation. Ce sont les associations de solidarité qui voient leurs files d'attente s'allonger. Ce sont les maires qui alertent sur le décrochage des quartiers populaires. Ce sont les jeunes qui risquent de devenir une génération sacrifiée. L'explosion de la pauvreté est alarmante. Si la mesure que nous avons adoptée pour renforcer le dispositif Coluche et encourager la générosité des Français est bienvenue, elle ne saurait servir d'unique instrument de solidarité. Nous avons proposé, en vain, d'améliorer la prise en charge du chômage partiel, d'augmenter les minima sociaux et de les étendre aux jeunes de 18 à 25 ans. Mes chers collègues, mon groupe ne revendique pas le monopole du coeur, mais il aimerait que la solidarité soit bien plus centrale dans la réponse de notre pays à la crise. Très bien ! Il en va de même en matière de transition écologique. En cette Journée mondiale du climat, à quelques jours des cinq ans de la signature de l'accord de Paris, sommes-nous à la hauteur Pourquoi avoir convoqué la Convention citoyenne sur le climat, si c'est pour refuser ensuite de mettre en oeuvre la plupart de ses recommandations ? Cette crise est une occasion manquée de préparer une reprise plus sobre et de changer notre modèle de développement en mettant la lutte contre le réchauffement climatique au coeur de la relance. Malheureusement, le Gouvernement a refusé de faire de la conditionnalité écologique un impératif. Et je ne parle pas de la majorité sénatoriale, qui a considéré qu'un malus tout à fait symbolique sur les 2 % de véhicules les plus lourds était déjà une contrainte insupportable pour notre industrie automobile Sur la transition énergétique comme sur la solidarité, nous sommes donc en profond désaccord avec ce projet de loi de finances. Monsieur le ministre, mes chers collègues, tout au long de l'examen du budget, le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain a fait des propositions pour plus d'équité fiscale et de justice sociale. Chaque dépense supplémentaire que nous proposions dans le cadre du plan de relance était compensée par des recettes nouvelles. J'ai entendu tout au long de nos débats la droite sénatoriale réclamer des réductions d'impôts sans jamais adopter la moindre baisse de dépenses tout en se désolant du déficit et de la dette publique. Pour notre part, nous avons le souci de la cohérence et de la responsabilité. C'est pourquoi nous avons voté pour une contribution exceptionnelle sur les assurances. Très bien ! Le choix de creuser le déficit plutôt que de mettre à contribution ceux qui en ont les moyens n'est pas le nôtre. Nous entendons maintenant la petite musique des déclarations ministérielles « quoi qu'il en coûte » aurait vécu, et la réforme des retraites redeviendrait d'actualité. Faute de faire contribuer les plus riches et les acteurs économiques, aujourd'hui, il faudrait faire payer tous les Français, même les plus modestes, demain. Quelle perspective injuste ! et malgré quelques ajouts positifs du Sénat, nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce projet de budget. Le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain votera contre.

Je tiens également à saluer le président de la commission des finances, Claude Raynal, qui a su mener

aussi les quarante-sept rapporteurs spéciaux de la commission des finances, les quatre-vingts rapporteurs pour avis des autres commissions et les chefs de file des huit groupes politiques, qui ont contribué au débat tout au long de ces semaines. je voudrais vous remercier, monsieur le ministre, de votre présence assidue au cours de l'examen des articles de la première partie, des crédits de la mission « Plan de relance » et des articles non rattachés de la deuxième partie, ainsi que de vos réponses toujours précises

Votre solitude a parfois suscité notre sollicitude, que j'ai exprimée au Premier ministre. J'aurai aussi l'occasion de le rappeler directement de nouveau aux ministres concernés. Il y va de la qualité de la relation entre l'exécutif et le Parlement.

Malgré ces contraintes et l'introduction d'une nouvelle mission « Plan de relance », qui a suscité- et c'est bien normal -de longs et légitimes débats, nous avons pu respecter les délais, mais en siégeant trois samedis sur les

Dans la discussion générale, la parole est à M. Hervé Maurey, coauteur de la proposition de loi.

collègues, en tant que deuxième cosignataire de la proposition de loi relative à la gouvernance et à la performance des ports maritimes français, déposée par notre ancien collègue Michel Vaspart et de nombreux collègues des groupes Les Républicains et Union Centriste, il me revient d'ouvrir aujourd'hui nos débats. Avant toute chose, je souhaite saluer le travail de Michel Vaspart, son engagement et ses compétences reconnues sur les enjeux maritimes et portuaires, qui ont permis à la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable d'approfondir ce sujet et de formuler des propositions concrètes. des propositions concrètes. À sa demande, nous avons constitué en novembre 2019 la mission d'information relative à la gouvernance et à la performance des ports maritimes, dont il a été tout naturellement le rapporteur. Cette mission a été présidée par Martine Filleul, dont je salue également le travail et l'implication. L'ensemble de la mission a effectué un travail de grande qualité qui a, comme très souvent dans notre assemblée, transcendé les clivages politiques.

une trentaine d'auditions et une dizaine de déplacements dans des ports maritimes, en France mais aussi à l'étranger, notamment à Anvers et Rotterdam, ont été organisés. Seule la situation sanitaire a empêché un déplacement à Gênes.

Toutefois, cette crise a mis en exergue le caractère stratégique des infrastructures portuaires et des chaînes logistiques pour l'approvisionnement de la Nation. Ainsi, après une période difficile, les professionnels se sont mobilisés, et je salue leur engagement. Cette mobilisation a été prolongée par la signature de la charte d'engagement des acteurs des chaînes logistiques françaises, le 7 octobre dernier, sous l'égide du ministre des transports, que je salue, et de la ministre de la mer. Je tiens à mentionner l'implication des professionnels pour assurer un transport fiable et compétitif des marchandises et privilégier le passage des marchandises par les ports français, en encourageant le recours aux modes massifiés. Il faut maintenant que cela se traduise dans les faits. Le travail de contrôle de la mission d'information a donné lieu au dépôt de deux propositions de loi : celle déposée par Michel Vaspart, que nous examinons aujourd'hui, et celle déposée par Martine Filleul et plusieurs collègues du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Ces initiatives complémentaires démontrent l'importance du sujet et l'intérêt du travail mené. Grâce à ces initiatives législatives, nous pouvons débattre concrètement des solutions à mettre en oeuvre pour nos ports. La proposition de loi dont nous allons débattre traduit les dix propositions formulées dans le rapport de la mission et les quatre recommandations adressées au Gouvernement.

le travail de Martine Filleul ont permis d'enrichir ce texte, qui contient des mesures importantes en faveur de l'attractivité de la place portuaire française et du nécessaire verdissement dans lequel notre économie s'engage. dix-sept articles de la proposition de loi ont vocation à couvrir tous les enjeux auxquels nos ports sont confrontés. Ils doivent permettre d'avancer concrètement sur des questions essentielles et de répondre aux demandes formulées de longue date par de nombreux acteurs. Je souhaiterais insister sur trois points, qui rejoignent les constats de la mission d'information. Tout d'abord, nous manquons d'une stratégie de long terme et d'une définition claire de la vision de l'État sur nos ports maritimes. Malgré le caractère stratégique de nos ports et la place de la France, deuxième puissance maritime mondiale, qui dispose de trois façades maritimes, nous attendons encore et toujours la stratégie nationale portuaire du Gouvernement, annoncée en novembre 2017.

Dans ce rapport, nous nous inquiétions déjà des faibles performances des ports français, au regard des objectifs qui avaient présidé aux différentes réformes portuaires et en comparaison avec les autres ports européens. Près de deux ans plus tard, nous en sommes malheureusement au même point. Dans son adresse aux Français prononcée le 14 juin dernier, le Président de la République a évoqué la nécessité « [d'accélérer] notre stratégie maritime, nous qui sommes la deuxième puissance océanique mondiale Malheureusement, si les annonces présidentielles et gouvernementales vont dans le bon sens, elles ne sont suivies d'aucun effet. Il est donc grand temps, monsieur le ministre, que le Gouvernement dévoile sa stratégie et la mette en oeuvre. est d'autant plus nécessaire que les Chinois sont de plus en plus présents, dans le cadre des nouvelles routes de la soie. Leurs participations dans les ports européens concernent désormais seize terminaux dans treize ports, et 10 % du volume des échanges. Je partage les inquiétudes de Michel Vaspart, qui nous a souvent alertés sur ce sujet et nous a appelés à faire preuve de plus de clairvoyance et de moins de naïveté. Le second point sur lequel je souhaite insister porte sur la problématique du sous-investissement chronique des infrastructures d'accès aux grands ports maritimes. Michel Vaspart s'était alarmé de la situation d'un grand nombre de lignes capillaires fret : certaines voies empruntées pour l'acheminement des récoltes depuis les silos céréaliers sont dans un tel état qu'il est aujourd'hui envisagé d'abandonner le rail au profit de la route. constatons d'ailleurs une baisse tendancielle de la part du transport ferroviaire dans le transport intérieur de céréales, qui est passée de 10 % pour la campagne 2012-2013 à 6 % pour la campagne 2017-2018. À Rouen, premier port céréalier d'Europe de l'Ouest, la part modale du fer ne représente que 6,8 %. Cette situation n'est pas acceptable. L'augmentation de la trajectoire de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France (Afitf), fixée par la LOM, est aujourd'hui indispensable pour enrayer cette tendance. En tant que rapporteur spécial de la commission des finances sur le budget des transports, je continuerai à être vigilant sur le soutien apporté par l'État à ses grands ports maritimes. Je constate que l'État, dans le projet de loi de finances pour 2021, a respecté ses engagements pour compenser l'intégralité des charges de dragage. un signal positif, même s'il faudrait aller plus loin et parvenir à une prise en charge substantielle et pérenne de l'ensemble des dépenses non commerciales des grands ports maritimes. Tel est l'objet de l'article 7 de cette proposition de loi. Par ailleurs, le rapport de la mission d'information a déjà produit des effets, puisque le Gouvernement a prévu un soutien au développement du fret ferroviaire, ainsi que des crédits spécifiques dédiés au verdissement des ports dans le cadre du plan de relance. Toutefois, quand nous examinons dans le détail le plan de relance, les 175 millions d'euros prévus sur deux ans semblent insuffisants, d'autant plus qu'ils sont destinés à financer de très nombreuses mesures, comme le développement des infrastructures de report modal, l'électrification des quais et la création de points d'avitaillement. Certes, Certes, des cofinancements sont prévus, mais l'effort de l'État aurait pu être plus important pour donner un véritable avantage comparatif à nos ports en matière de transition écologique. Une augmentation de l'aide à la pince est également prévue, mais elle reste insuffisante par rapport aux 80 millions d'euros proposés par la mission qui, seuls, pourront permettre de restaurer la compétitivité du transport combiné intérieur. Le plan de relance n'est donc pas aussi ambitieux que les propositions de la mission d'information. Il constitue un premier pas positif, qui nécessite cependant Avant de conclure, je forme le voeu que la vie de cette proposition de loi se poursuive au-delà de son examen par le Sénat, et qu'elle puisse également être discutée à l'Assemblée nationale.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons cet après-midi a été déposée le 24 septembre dernier par notre ancien collègue Michel Vaspart et de nombreux autres sénateurs. dix-sept articles de ce texte et son rapport annexé renvoient fidèlement aux propositions de la mission d'information présidée par Martine Filleul, que je salue, et dont le rapporteur était Michel Vaspart. Cette mission avait été mise en place par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable en novembre 2019. Je souhaite, à mon tour, rendre un hommage particulier à notre ancien collègue et mon ami Michel Vaspart pour son implication et son travail sur ces sujets. Le rapport de la mission d'information a été adopté à l'unanimité en commission le 1 juillet dernier témoigne de l'importance du travail réalisé et de l'attention portée à ce sujet par tous les groupes politiques de notre assemblée. Je ne reviendrai pas sur les constats, qui sont connus. Près de vingt rapports ont été écrits sur nos ports depuis dix ans, soit deux par an en moyenne, dont la plupart à la demande du Gouvernement. Pourquoi sommes-nous ici aujourd'hui ? S'il est vrai que le secteur portuaire a fait l'objet de réformes de grande ampleur depuis le début des années 1990, qui ont permis à nos ports, en particulier aux grands ports maritimes relevant de l'État, de redresser leurs finances et leur compétitivité, leurs performances demeurent décevantes. Les faits en attestent. Au total, en 2020, le trafic des sept grands ports maritimes métropolitains est inférieur de plus de 40 % à celui du seul port de Rotterdam, par lequel transite également un tonnage trois fois plus important de conteneurs. plus important de conteneurs. Plus de 40 % des conteneurs à destination de la France métropolitaine transitent encore aujourd'hui par des ports étrangers. Le retard accumulé par la France est tel que nous estimons qu'entre 30 000 et 70 000 emplois seraient perdus. Dans les documents annexés au projet de loi de finances pour 2021, le Gouvernement a révisé la prévision de part de marché des grands ports maritimes de 13 % à 12,5 % pour 2020, par rapport aux trente-deux ports européens pris pour référence, avec une part de marché de la filière des conteneurs qui pourrait s'établir à 6,1 % au lieu de 6,5 % pour 2020.

dans le transport massifié de marchandises, ainsi que d'une image de fiabilité encore écornée auprès des grands chargeurs et armateurs. La proposition de loi prévoit d'ailleurs de dégager davantage de moyens en faveur de la massification des acheminements portuaires. Sans politique ambitieuse de massification du transport de marchandises, il est illusoire d'imaginer que nos ports gagnent durablement des parts de marché, alors que, dans le même temps, 50 % du fret en conteneurs du port d'Hambourg est acheminé par voie ferroviaire ou fluviale.

Une augmentation conséquente de la trajectoire d'investissement de l'Afitf, fixée par la LOM, est indispensable pour parvenir véritablement à renforcer la compétitivité de nos ports. À ces éléments de compétitivité hors prix s'ajoute le principal constat de notre commission, à savoir une absence de vision stratégique à long terme de l'État sur nos ports, à cette date. Vous nous indiquerez sans doute, monsieur le ministre, à quel moment sera présentée la stratégie nationale portuaire. La création d'un Conseil national portuaire et logistique (CNPL) et l'inscription dans le code des transports de la stratégie nationale portuaire, prévues par l'article 1 de la proposition de loi, répondent à ce besoin qui a d'ailleurs été relevé par la quasi-totalité des acteurs que j'ai consultés, ainsi que par Michel Vaspart et la mission. Certes, monsieur le ministre, un Comité France maritime (CFM) étoffé existe déjà, mais aucune des instances existantes ne présente un caractère transversal, permettant d'associer à la fois le côté mer et le côté terre, en prenant en compte l'ensemble des acteurs de la chaîne portuaire et logistique. En outre, le CNPL n'a pas été conçu comme un arbre de plus dans la forêt des instances placées auprès du Gouvernement. Il a vocation à intégrer des structures existantes, dont certaines sont pour l'heure peu dynamiques, comme l'Observatoire des coûts de passage portuaire ou encore le comité interministériel de la logistique (Cilog), même si ce dernier s'est réuni hier avec des ambitions affichées. C'est une logique de rationalisation et non de complexification qui répond à cette volonté de création du CNPL. Nos concurrents européens et internationaux sont mieux organisés que nous. La stratégie portuaire et logistique allemande fait l'objet d'un débat au Bundestag et figure dans le contrat de coalition du gouvernement actuel. Les Britanniques, malgré la privatisation de leurs ports en 1986, ont maintenu un travail de prospective. Surtout, la République populaire de Chine a lancé une initiative d'une ampleur peu commune, avec les nouvelles routes de la soie, qui incluent évidemment une dimension maritime. Michel Vaspart était et reste particulièrement préoccupé par ce sujet, comme nous tous. Il a alerté plusieurs ministres depuis deux ans. Quand nous interrogeons les administrations de l'État sur les évolutions apportées pour la protection de nos actifs stratégiques et le contrôle des investissements étrangers, c'est tout juste si l'on ne nous répond qu'il n'y a pas de problème et que tout est sous contrôle. Les seuils de contrôle des investissements étrangers ont été temporairement abaissés jusqu'au 31 décembre 2020. Dont acte. Je doute que cela soit suffisant. Vous nous parlerez sans doute des discussions que vous menez à l'échelle de l'Union européenne. Je constate que l'information du Parlement et des élus nationaux sur ces sujets est trop faible, alors que nous pourrions un jour être amenés à voter des dispositions en la matière si la situation évoluait défavorablement pour certaines de nos entreprises. Le rapport de notre commission a également mis en lumière des frustrations et des incompréhensions issues des réformes de 2008 et 2016, qui ont conduit à l'exclusion des acteurs économiques des instances décisionnaires des ports, au nom de la prévention des conflits d'intérêts. Pourtant, des outils de prévention et de gestion des conflits d'intérêts existent, y compris dans le code des transports. Il serait bon de les utiliser de manière pragmatique, plutôt que de refuser par principe toute association ou implication du secteur privé.

représentatives de la diversité des parties prenantes et placées en situation d'exercer un réel contrôle de la direction de l'établissement. Au-delà, l'avenir de nos ports est étroitement lié à celui du modèle économique du transport de marchandises, et plus largement à la structure de notre économie, fortement importatrice- nous pouvons évidemment le regretter. Nos ports se retrouvent pris en étau entre la baisse de leurs recettes, liées en particulier au trafic d'hydrocarbures, et la hausse de leurs charges non commerciales et fiscales- Je resterai donc attentif à la mise en oeuvre des mesures votées dans le cadre du projet de loi de finances pour 2021. Avant de conclure, je rappellerai les trois principaux axes de travail retenus en commission sur ce texte. Le premier axe renforcer l'intégration des collectivités territoriales à la politique portuaire, pour favoriser la coordination entre l'ensemble des ports, associer avec discernement et mesure les acteurs privés à la gouvernance des établissements portuaires, et ainsi améliorer à la marge le cadre issu des lois de 2008 et 2016. J'ai mené le travail préparatoire à l'examen de cette proposition de loi dans le souci de préserver les propositions de Michel Vaspart, mais en y apportant des ajustements et des compléments sur des sujets ponctuels.

deuxième axe est d'améliorer l'attractivité et la compétitivité de nos grands ports maritimes et des ports des collectivités territoriales. La commission a notamment adopté deux amendements visant à créer des zones de relance économique temporaires et un dispositif de suramortissement, pour favoriser les investissements concourant à la fluidité du passage portuaire, avec une double conditionnalité sectorielle et environnementale. Enfin, le troisième axe est de soutenir le verdissement de ce secteur, en offrant des outils supplémentaires aux acteurs pour les accompagner activement dans la transition écologique. Vous le voyez, monsieur le ministre, nous sommes mobilisés pour soutenir nos ports et la relance de l'économie. Nous sommes prêts à y travailler avec vous et avec nos collègues députés. Je Je terminerai par une question très simple, qui rejoint celle posée par Hervé Maurey en conclusion de son propos : le Gouvernement va-t-il se décider à saisir cette proposition que nous lui faisons ? Je vous remercie monsieur le ministre, « Homme libre, toujours tu chériras la mer ! », tel était le commandement de Charles Baudelaire. Aujourd'hui, chérir la mer exige de chérir les portes qui nous y mènent. Ces portes, ce sont nos ports. Notre ambition est de les rendre plus forts, tant en matière de gouvernance que de performance. Telle est l'ambition du Gouvernement. C'était hier celle du rédacteur de cette proposition de loi, Michel Vaspart, qui a longtemps siégé sur ces travées. C'est aujourd'hui la vôtre, madame la présidente de la mission d'information, monsieur le rapporteur et monsieur le premier signataire de fait, cher Hervé Maurey. Je sais combien la puissance maritime de la France importe au Sénat. Je sais combien vous êtes attachés à ce que notre pays tire pleinement profit de ses grandes façades maritimes et de ses nombreux territoires ultramarins. Cet attachement, cette attention, ces égards qui sont les vôtres, je les retrouve dans le texte que nous allons examiner. Toutefois, celui-ci a été rédigé dans un contexte bien différent. Depuis, la crise sanitaire a frappé le monde. Le Gouvernement a très rapidement pris des engagements, qui ont d'ores et déjà défini les jalons de notre stratégie maritime. Dès cet été, le Président de la République en a présenté les grandes lignes. En septembre, avec le plan de relance, nous avons annoncé des investissements massifs, dont 400 millions d'euros dédiés aux secteurs maritime et fluvial- leur avenir doit en effet être pensé de pair -, et 1 milliard d'euros en faveur du fret ferroviaire qui permettra, notamment, la création d'autoroutes ferroviaires reliant plusieurs ports entre eux. En octobre, nous avons signé la charte portuaire. Elle contient des engagements clairs et inédits de la part des acteurs de la filière logistique, des donneurs d'ordre et des partenaires sociaux. En novembre, nous avons nommé un directeur général préfigurateur pour Haropa ports de Paris Seine Normandie, et les discussions se poursuivent pour approfondir ce projet portuaire majeur. Nous avançons, mais nous n'allons pas nous arrêter là.

premier mot d'ordre est donc de renforcer la compétitivité de nos ports. Cela passe par un coût de passage portuaire optimisé. À cet effet, nous expérimentons le point de contact unique aux frontières, au Havre, à Marseille et à Dunkerque. La compétitivité passe aussi par un dialogue social de qualité, pour prévenir les conflits et ainsi conférer à nos ports davantage de fiabilité. C'est tout l'objet de la charte portuaire signée en octobre par les acteurs des chaînes logistiques et des filières maritime, portuaire, fluviale et ferroviaire françaises. La compétitivité passe également par la reconquête des parts de marché. Pour la mener à bien, nous devons faire de nos ports des maillons plus solides d'une chaîne logistique véritablement intermodale. Cela implique de renforcer l'intermodalité et d'accroître le report modal vers les transports massifiés, alors que, aujourd'hui, la part du fret vers ou depuis la France qui est manutentionnée dans les ports français est d'environ 60 %. Notre objectif est de la porter à 80 % d'ici à 2050. Nous devons mettre nos ports au service de la relance des territoires. Il nous faut, pour cela, favoriser l'implantation de nouveaux industriels et logisticiens dans les zones industrialo-portuaires. Notre objectif, à l'horizon de 2050, est de doubler le nombre d'emplois directs et induits liés à l'activité portuaire.

Cet objectif de reconquête sera au coeur de la stratégie nationale portuaire. Elle sera présentée au début de l'année prochaine, à l'occasion du comité interministériel de la mer (CIMer). J'en suivrai personnellement la mise en oeuvre, en lien avec la ministre de la mer et les différentes parties prenantes.

Des outils de souveraineté ont été renforcés par le Gouvernement. Il faut les utiliser lorsque cela est nécessaire- je pense notamment au décret relatif aux investissements étrangers en France. Notre souveraineté dépend aussi de la bonne coordination entre nos ports d'État et nos ports décentralisés, et entre nos ports maritimes et intérieurs. Face à des alliances maritimes très puissantes, elle est indispensable. Les travaux se poursuivent au sein des axes logistiques et portuaires pour renforcer cette souveraineté, et accroître l'hinterland des ports français le long des axes fluviaux et ferroviaires. Les enjeux d'intermodalité sont cruciaux en la matière. La souveraineté donne aussi son sens à l'intégration des ports du Havre, de Rouen et de Paris, qui sera effective d'ici à l'été 2021. Avec Haropa, nous sommes en train de bâtir une porte d'entrée unifiée pour le premier ensemble portuaire français, un ensemble capable de rivaliser avec ses principaux concurrents européens. Si, au vu de son intérêt stratégique pour la Nation, il a vocation à demeurer sous contrôle de l'État, il associera fortement les collectivités qui seront parties prenantes à sa gouvernance. Un directeur général préfigurateur a été nommé en la personne de Stéphane Raison. Il a pour mission de mener à bien la finalisation du processus de fusion, en s'appuyant sur les travaux menés par Catherine Rivoallon.

le plan de relance, avec 175 millions d'euros sur deux ans qui iront aux grands ports maritimes de métropole et d'outre-mer, et aux ports autonomes de Paris et Strasbourg. Ils permettront, par exemple, d'accélérer la modernisation de l'écluse de Tancarville au Havre, ou encore l'électrification des quais croisière et ferries à Marseille. Nous soutiendrons également les investissements des collectivités en faveur des ports décentralisés, la dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). Nous en avons triplé le montant annuel en juin dernier, et les ports y sont éligibles. Monsieur le rapporteur, vous pouvez le constater, le Gouvernement agit pour rendre nos ports plus forts, plus durables. Nous partageons de nombreuses idées contenues dans cette proposition de loi, à tel point que nous sommes déjà en train de les mettre en oeuvre. ce vecteur législatif est-il adapté, alors que nombre de ces mesures sont de nature réglementaire, que certaines sont déjà en vigueur et que d'autres sont à approfondir en concertation avec les territoires et les partenaires sociaux ? Je ne le pense pas. Pour autant, je tiens à ce que nous puissions travailler de concert, sur plusieurs sujets. Je pense, tout d'abord, à la meilleure inclusion des parlementaires dans nos comités de pilotage et de suivi, comme celui qui résultera de la mise en place de la stratégie nationale portuaire, plutôt qu'à la création de nouvelles instances. Je pense aussi à l'opportunité de venir plus régulièrement rendre compte de notre action dans cet hémicycle, sans que cela soit inscrit dans la loi, lors d'une mise à jour de la stratégie tous les cinq ans. Tel est le sens de l'article 1 de la proposition de loi. Nous y répondrons en janvier. Je pense, par ailleurs, à la mise en place de contrats pluriannuels d'objectifs et de performance (COP) entre l'État et les ports. Tel est le sens de l'article 7 de votre proposition de loi. Nous allons approfondir cette mesure avec mes services. services. Le plan de relance nous permet d'investir davantage dans le verdissement du secteur. Nous approuvons ainsi en grande partie les articles 13 et 14. Trouvons ensemble les moyens d'une meilleure communication, afin que ces crédits permettent de soutenir des projets stratégiques pour nos ports. Voilà les sujets sur lesquels je vous propose de travailler, à l'issue de nos débats et hors cadre législatif. Néanmoins, nous ne sommes pas d'accord sur tout. Je souhaite m'arrêter sur trois sujets, sur lesquels des divergences sont à noter. Car l'enjeu pour nos ports est moins d'engager une nouvelle évolution de leur gouvernance ou une nouvelle étape de leur décentralisation, que de les aider à reconquérir des parts de marché. Sur le sujet de leur gouvernance, le texte que nous examinons modifierait fortement les équilibres issus de la réforme portuaire de 2008 et de la loi pour l'économie bleue de 2016. Certaines mesures s'inscrivent même à rebours de l'esprit de la réforme de 2008, qui a pourtant montré son efficacité. Dans le contexte d'une intense concurrence européenne et mondiale, il n'est pas certain que cette proposition de loi aille dans le sens d'une meilleure compétitivité, d'une bonne coordination nationale et d'une reconquête des parts de marché. Elle pourrait même constituer un facteur d'instabilité supplémentaire. Sur le sujet de la décentralisation des ports, le texte ouvrirait cette possibilité aux régions qui en feraient la demande. Toutefois, aucune des régions avec lesquelles l'État a pu engager une réflexion ne le demande. En outre, les grands ports maritimes qui, après les différentes étapes de la décentralisation, demeurent aujourd'hui sous contrôle de l'État, sont soit d'un intérêt stratégique pour la Nation, car ce sont des portes d'entrée sur notre territoire, soit des ports ultramarins, essentiels à la continuité territoriale. C'est pourquoi la conviction du Gouvernement est que l'État doit en garder la responsabilité, en lien étroit avec les collectivités. J'entends néanmoins, de la part des présidents de région, que l'État doit pouvoir garantir un soutien sans faille aux trajectoires d'investissement de chaque grand port d'État. C'est bien l'ambition du Gouvernement, et cela va se traduire dans les négociations budgétaires en cours, pour les territoires concernés, dans le cadre de l'élaboration des nouveaux contrats de plan État-région Enfin, concernant les services portuaires, les dispositions que vous proposez pourraient conduire à imposer un service minimum. Leur application poserait des difficultés majeures, et tout d'abord des difficultés juridiques, car cela reviendrait à réquisitionner des personnels d'entreprises privées

La signature de la charte portuaire a permis de poser les bases durables d'un climat social apaisé dans les ports français, indispensable à la continuité de leur activité. Nous souhaitons poursuivre dans cette voie, en fonctionnant en, comme au rugby, avec la communauté portuaire.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous demanderai de considérer que c'est mon collègue Ronan Dantec, cloué au lit par la fièvre, qui s'exprime par ma voix. Les grands ports maritimes sont à la croisée des enjeux économiques, sociaux et environnementaux des territoires. En tant qu'écologistes, nous sommes extrêmement soucieux du devenir des ports. le transport maritime constitue à nos yeux une alternative majeure au transport routier et il faut qu'il contribue, lui aussi, à une économie décarbonée. L'avenir des grands ports maritimes se trouve à une période charnière. Nous avons pris du retard nous attendons la stratégie nationale portuaire annoncée depuis 2017 par le Gouvernement. Le texte que nous examinons aujourd'hui est donc bienvenu.

en particulier les grands ports maritimes relevant de l'État, têtes de pont et premières portes d'entrée du commerce extérieur français », qui sont concurrencés par les ports de la mer du Nord. Il prévoit la création d'un Conseil national portuaire et logistique (CNPL), l'implication des acteurs économiques et locaux dans la gouvernance, davantage de décentralisation sur demande, l'institution d'un contrat de compétitivité et d'objectifs, et enfin le verdissement des ports. En avril 2018, l'Organisation maritime internationale (OMI) a pour la première fois adopté une stratégie de décarbonation ambitieuse, avec un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'au moins 50 % à l'horizon 2050 par rapport à 2008, et un objectif intermédiaire de réduction d'au moins 40 % d'ici à 2030. Je tiens à rappeler que le Sénat avait voté, lors de l'examen du projet de loi d'orientation des mobilités, l'inscription législative de la stratégie de transition énergétique concernant le transport maritime-

Cet article dispose également que l'État doit engager « une concertation avec l'ensemble des parties prenantes afin de définir une stratégie visant à accélérer la transition vers une propulsion neutre en carbone à l'horizon 2050 pour l'ensemble des flottes de commerce, de transport de passagers, de pêche et de plaisance sous pavillon national. » Monsieur La décarbonation du transport maritime passe, par exemple, par le développement des raccordements électriques à quai qui permet de limiter la production de pollution sur le lieu d'accostage. C'est l'objet de la proposition SD-B2.2 « Électrification des quais » de la Convention citoyenne pour le climat, que le Gouvernement considère avoir déjà mis en oeuvre les 175 millions d'euros du plan France Relance et les lois de finances rectificatives pour 2020. Nous serons vigilants sur ce point ! Il est, à cet égard, bienvenu que les articles 13, 14 et 15 de cette proposition de loi renforcent les moyens du verdissement. Le plan de relance insiste aussi beaucoup sur l'hydrogène concernant la motorisation. Nous sommes inquiets de l'absence de précision sur le ferroviaire, sur la question du ferroutage et des liaisons ferroviaires et fluviales au départ des grands ports maritimes. J'espère, monsieur le ministre, que la discussion permettra de préciser les investissements que vous avez prévus dans ce domaine, les liaisons ferroviaires au départ des ports maritimes étant la faiblesse structurelle des ports français pour leur compétitivité.

Il est question de créer un parc écotechnologique dédié aux énergies marines renouvelables, mais nous ne savons pas à ce stade avec quelles entreprises. L'absence de réponse des autorités portuaires aux interrogations des collectivités territoriales qui ont exprimé leur scepticisme dit clairement l'impasse qui existe aujourd'hui sur la question de la gouvernance des ports. Il faut que les élus locaux et régionaux soient mieux informés et associés, et la régionalisation de certains grands ports ne doit pas être un tabou. Derrière cette régionalisation, il y aura aussi le dialogue entre les ports. Le développement du transport maritime, ce n'est pas uniquement une question de « grands » ports, car il faut une articulation entre les différents types de ports et de liaisons, y compris le cabotage. Nous restons convaincus de l'importance du cabotage, qui renforcerait les petits ports. Soulignons également l'importance du transport combiné entre le transport maritime et le transport fluvial, qui nécessite des créations d'emplois de dockers et de manutentionnaires.

nous partageons l'ambition de renforcer l'attractivité de nos ports et d'augmenter leurs parts de marché. Il nous faut ni plus ni moins bâtir les infrastructures du XXI siècle. Cette proposition de loi a été déposée par un parlementaire breton, M. Vaspart, ancien sénateur des Côtes-d'Armor. Elle fait suite à la mission d'information qui était présidée par Mme Filleul Nous saluons le travail ainsi accompli sur un sujet fondamental, alors que la France a un accès à tous les océans et qu'elle possède le deuxième plus grand domaine maritime du monde. Une trentaine d'auditions et une dizaine de déplacements ont été organisés pour établir un état des lieux en matière de compétitivité, avec trois angles d'approche : la gouvernance, le volet social et l'aménagement du territoire.

dans les stratégies de développement portuaire. Au regard de la crise sanitaire, du Brexit et des transformations écologiques, économiques et technologiques, un nouvel élan est aujourd'hui indispensable. Quel est le constat ? Les trafics dans les grands ports maritimes ont reculé depuis douze ans ; le niveau est revenu à celui d'il y a vingt ans. Les coûts de passage portuaire sont plus élevés que ceux de nos concurrents. un sous-investissement chronique dans les infrastructures. Il nous faut enfin constater une insuffisance de notre système logistique. Je fais d'ailleurs écho ici à mon propos préalable : à l'heure actuelle, nos acheminements portuaires reposent toujours en grande partie sur le mode routier, routier, alors que d'autres solutions, ferroviaires et fluviales, devraient être possibles. Soulignons enfin que 40 % des conteneurs à destination de la France métropolitaine transitent encore par des ports étrangers. Ce sont des dizaines de milliers d'emplois qui partir de ce diagnostic partagé, je me permets de vous soumettre quelques interrogations sur la traduction législative. Sur le calendrier, tout d'abord, la stratégie nationale portuaire sera présentée prochainement de la mer, s'est engagée à ce que cette feuille de route soit présentée avant le prochain comité interministériel de la mer afin de convertir, dans les années à venir, notre potentiel de croissance.

Rappelons que le plan de relance, dont nous avons récemment discuté, prévoit 200 millions d'euros en autorisations d'engagement pour le verdissement des ports et de la flotte des affaires maritimes. En outre, nous ne sommes pas favorables à l'article 8 qui porte sur la disponibilité des services portuaires, en particulier du remorquage. Nous ne minimisons pas le sujet, mais il nous semble tout aussi capital de pacifier le dialogue social. Alors que ce dispositif reviendrait à instaurer un service minimum, les organisations syndicales doivent être associées à nos débats. Sans compter les problèmes d'ordre juridique qui découleraient d'une telle disposition. Nous nous interrogeons aussi sur le processus de régionalisation des grands ports maritimes, proposé à l'article 6 : est-ce une priorité aujourd'hui et sous cette forme ? Nous craignons enfin que la création d'un nouveau Conseil, en plus du Conseil supérieur de la marine marchande (CSMM), ne fasse doublon et n'ajoute de la complexité. En conclusion, je voudrais attirer l'attention sur les grands ports, mais aussi sur les moins grands, ceux qui ne sont pas classés « grands ports maritimes » et qui devront être pleinement intégrés dans la stratégie nationale à venir. J'évoquerai les ports bretons- vous avez compris que j'étais Bretonne ! -, celui de Brest en particulier, qui constituent un maillon essentiel de nos politiques de transport. Ils font pleinement partie du réseau national et accueillent de nombreuses activités, logistiques et touristiques, industrielles et de réparation navale. Le renforcement de leur compétitivité est également indispensable, comme leurs responsables le réclament. Si nous saluons le débat rendu possible par ce texte,

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, presque trente ans se sont écoulés sans que la France, qui détient pourtant la deuxième superficie maritime au monde avec 11 millions de kilomètres carrés de zone économique exclusive (ZEE), dispose d'un ministère de la mer de plein exercice. Est-ce un tournant ? Je l'espère, monsieur le ministre, car l'heure est grave pour notre économie maritime, structurellement fragilisée et frappée, elle aussi, par la crise sanitaire. Je tiens à remercier notre ancien collègue Michel Vaspart et les membres de la mission d'information présidée par Martine Filleul, qui ont réalisé un travail considérable et riche de recommandations, lesquelles ont été reprises par la présente proposition de loi et complétées judicieusement en commission.

Cet article permettra à l'ensemble des acteurs d'être associés à l'élaboration de la politique maritime, et au nouveau Conseil national portuaire et logistique de vérifier que la trajectoire des investissements est cohérente avec la stratégie. Si les responsabilités des échecs de la politique maritime ne peuvent être exclusivement attribuées à la gouvernance des ports, des modifications législatives à la marge peuvent néanmoins contribuer à instaurer un dialogue plus efficace entre les instances. La coopération à tous les niveaux est en effet la clé de la compétitivité. Nous saluons ainsi la réduction du nombre de membres siégeant au sein du conseil de surveillance, l'attribution de sa présidence à un représentant des collectivités territoriales et l'intégration du président du conseil de développement. Nous proposons néanmoins un amendement visant à réintégrer la nomination d'un représentant de la chambre de commerce et d'industrie (CCI). Par voie d'amendement, nous proposons également de renforcer le dialogue entre le conseil de développement, par la voix de son président, et le conseil de surveillance. Enfin, la mise en place de contrats pluriannuels d'objectifs et de performance ou encore la révision de la procédure de révocation du directeur général oriente la politique portuaire vers l'obtention de résultats, ce qui est de nature à nous rassurer. Nous sommes conscients que le sujet relatif à la décentralisation des ports divise- c'est d'ailleurs le cas au sein de mon groupe. S'il convient de laisser aux régions le choix de se saisir de cette compétence, il incombe à l'État de donner ou non son accord pour des raisons stratégiques, en lien avec les intérêts européens et internationaux.

préserverait l'exercice des missions régaliennes par l'État et apporterait le bénéfice d'une vision stratégique territorialisée. Pour reprendre les mots prononcés lors des Assises de l'économie de la mer de 2017 par Édouard Philippe, alors Premier ministre : « L'échelon pertinent, c'est la région.

trafic de conteneurs. La LOM a constitué une occasion manquée d'accélérer sur ce dossier, alors que- nous en sommes convaincus -le grand port maritime de Bordeaux recèle un potentiel d'innovation certain, comme en témoigne l'obtention en juillet dernier d'un appel à projets européen visant à déployer l'hydrogène en milieu portuaire en tant que carburant alternatif. Afin de renforcer l'attractivité de nos ports, la commission a introduit des mesures que nous jugeons pertinentes, telles que l'institution de zones de relance économique temporaires bénéficiant d'un régime douanier et fiscal venant soutenir l'implantation d'activités à haute valeur ajoutée industrielle, conditionné au respect d'exigences environnementales. de même pour le dispositif de suramortissement des biens, équipements, matériels et technologies améliorant la fluidité du passage portuaire et la chaîne logistique ou réduisant les émissions polluantes, tout en participant pleinement à la modernisation et à la transformation écologique du secteur portuaire. Les grands ports maritimes ne gagneront pas en compétitivité sans le développement de l'hinterland. Prévu par le rapport annexé à la proposition de loi, le doublement des moyens consacrés au report modal vers les transports ferroviaire et fluvial, pour atteindre 5 milliards d'euros sur dix ans, est à ce titre indispensable pour rattraper le retard que nous avons pris par rapport à nos voisins européens. Au regard des avancées proposées par ce texte, la grande majorité du groupe RDSE le soutiendra. La parole

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi qui nous est soumise résulte d'une mission d'information de notre assemblée et je voudrais, à mon tour, saluer l'engagement de Michel Vaspart, sénateur des Côtes-d'Armor. La Bretagne,

cherche sa place dans le vaste concert mondial et nourrit quelques ambitions en matière de développement de ses petits ports. Le premier mérite de cette initiative parlementaire est d'affirmer que notre pays a besoin d'une grande ambition portuaire et maritime, et que cette ambition appelle une grande volonté politique. Vous l'avez rappelé, monsieur le ministre- dont acte

Le texte met en avant certaines orientations, notamment la nécessité d'investissements sur les liaisons entre les ports, et avec leur hinterland et l'ensemble du territoire. On peut considérer que les ports ont deux grandes missions une mission publique de développement du territoire- nul besoin de développer tout ce que cela implique -et une mission marchande, avec laquelle il convient de composer. Pour véritablement changer la donne, il conviendrait d'avoir une grande ambition publique pour la mission publique,

consisterait à permettre aux ports de tenir un double bilan financier avec un budget fourni par la tutelle publique pour les missions publiques et un bilan de type privé pour les missions marchandes, en prévoyant que les privés participent au financement des missions marchandes. Il n'en est pas vraiment question dans la proposition on me rétorquera peut-être que les ports déjà décentralisés pourraient trouver leur place dans un projet construit exclusivement autour des Peut-être ! Mais je vous avoue que cela me trouble : en effet, par extension de ce même raisonnement aux politiques terrestres, on pourrait aussi suggérer que nos petits territoires n'auraient plus qu'à rechercher leur place dans les espaces configurés et laissés libres

Ce texte vise à créer un cadre propice à la reconquête de parts de marché pour nos ports maritimes, en particulier les grands ports maritimes relevant de l'État, premières portes d'entrée du commerce extérieur français. Il faut savoir que 90 % des échanges mondiaux se font par voie maritime. Autant dire que les ports français sont des acteurs stratégiques dans ce domaine, avec un impact économique considérable. La valeur ajoutée du fonctionnement du système portuaire français dépasse les 15 milliards d'euros et l'activité portuaire représente plus de 350 000 emplois directs et indirects. La France possède de nombreux points forts, avec ses trois façades maritimes métropolitaines, son accès à tous les océans grâce à l'outre-mer, son deuxième plus grand domaine maritime au monde et son dense réseau de soixante-six ports de commerce.

Nos ports maritimes sont aujourd'hui confrontés à une forte mutation du transport maritime : augmentation de la taille des navires, concentration économique, numérisation et reconfiguration du paysage géopolitique, avec notamment la mise en oeuvre de la stratégie chinoise des nouvelles routes de la soie.

Ce constat terrible, j'ai aussi dû le relire plusieurs fois ! De nouvelles stratégies de reconquête s'avèrent donc nécessaires pour valoriser ce domaine essentiel à l'économie française. Les potentialités de croissance sont très importantes, y compris à court et moyen termes. Ces mesures pourraient représenter une hausse de 10 % de la part de marché des grands ports maritimes sur le trafic de conteneurs, associée à plus d'un milliard d'euros de valeur ajoutée, ainsi qu'à la création de 25 000 emplois directs et indirects. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui reprend les mesures proposées par la mission d'information relative à la gouvernance et à la performance des ports maritimes. Bien sûr, on est en droit de s'interroger sur la nature de ce véhicule législatif pour aborder des sujets aussi stratégiques. Néanmoins, l'intention est là et cette proposition de loi tend à moderniser et améliorer la gouvernance des ports français, en instituant une stratégie nationale portuaire et en créant un Conseil national portuaire et logistique chargé du suivi de sa mise en oeuvre. Ce CNPL renforcerait la représentation des collectivités territoriales et des acteurs économiques de la place portuaire au sein du conseil de surveillance de chaque grand port maritime. Cette proposition de loi tend également à renforcer les pouvoirs du conseil de développement des grands ports maritimes, en leur permettant de rendre un avis conforme sur le projet stratégique de l'établissement. Elle comporte aussi des mesures visant à clarifier le fonctionnement des conseils de coordination interportuaire. Ce texte vise également à renforcer l'attractivité et la compétitivité des grands ports maritimes, en favorisant leur développement, notamment grâce à des mesures relatives à l'exécution et à la régulation des services portuaires de pilotage et de remorquage. Nous ne pouvons que soutenir l'ensemble de ces orientations, qui vont dans le bon sens, d'autant que le texte a été notablement amélioré par les travaux de notre commission de l'aménagement du territoire et du développement durable, qui a assoupli les modalités de gouvernance et qui est parvenue à une meilleure représentation de l'ensemble des acteurs concernés. La commission a aussi renforcé la compétitivité et le verdissement du secteur. Elle propose notamment d'instituer des zones de relance économique temporaires, avec un régime douanier et fiscal spécifique, et de définir un régime de suramortissement à hauteur de 30 % pour l'acquisition de certains équipements et technologies concourant à la fluidité du passage portuaire et de la chaîne logistique. Accompagner la transition écologique de ce secteur a également été, je vous l'ai dit, une priorité de nos travaux en commission. Des outils incitatifs ont été mis en place pour que les acteurs du domaine portuaire s'engagent clairement et plus fortement à réduire leur impact environnemental. Le mécanisme de suramortissement que je viens de citer vise notamment l'acquisition d'équipements permettant une réduction d'au moins 25 % des émissions de CO2, de soufre ou de tout type de pollution. La commission a également souhaité ouvrir la possibilité pour les grands ports maritimes volontaires d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan d'optimisation des coûts et, le cas échéant, de réduction du surcoût de manutention fluviale, afin de favoriser le report modal et le verdissement du transport de marchandises. Ces différentes mesures doivent permettre une relance économique verte de nos ports maritimes français. Un mot maintenant de la mesure sur laquelle vont sans doute se concentrer nos débats débats : le fameux article 6, qui ouvre la possibilité d'une décentralisation de la propriété, de l'aménagement, de l'entretien et de la gestion des grands ports maritimes aux régions qui en feraient la demande, sous réserve de l'accord de l'État. Pour ma part, autant la possibilité d'une telle décentralisation me semble judicieuse pour la gestion des ports intérieurs, autant j'entends les arguments de ceux qui considèrent que cette décentralisation risquerait de mettre à mal la stratégie nationale. Les débats que nous aurons dans cet hémicycle nous permettront probablement d'obtenir des éclairages très intéressants. Quoi qu'il en soit, la présente proposition de loi est de nature à créer un écosystème portuaire en phase avec nombre de priorités pour l'aménagement des territoires, comme la réalisation concomitante du barreau nord-est et du barreau sud-est pour le contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise, ou le triplement de l'aide à la pince afin de soutenir le report modal. Je pense aussi, bien sûr, au développement de plateformes logistiques le long de l'attendu canal Seine-Nord Europe. Ce projet, que je connais bien pour en être l'ambassadeur depuis plus de vingt-cinq ans, d'abord à la région, puis à l'Assemblée nationale et dorénavant au Sénat, avec mon collègue Laurent Somon ici présent, est un projet majeur qui constituera un maillon central de la liaison fluviale européenne à grand gabarit Seine-Escaut. En reliant les bassins de la Seine et de l'Oise aux 20 000 kilomètres de réseau fluvial nord-européen à grand gabarit, il permettra de faire voguer des bateaux de fret fluvial de 4 400 tonnes, soit l'équivalent de deux cent Ce report modal de la route vers la voie d'eau entraînera une diminution importante des émissions de CO2, décongestionnera les autoroutes de l'axe concerné et surtout créera des milliers d'emplois conjoncturels, le temps des travaux, et structurels grâce aux plateformes d'irrigation économique le long de son parcours. C'était mon couplet picard ou plus exactement, madame la présidente, mon couplet haut-français ... Vous l'aurez compris, il nous semble urgent de donner un nouvel élan à nos ports maritimes français, de renforcer leur compétitivité et de soutenir leur verdissement. Sceptique quant à la durée de vie de cette proposition de loi, le groupe Union Centriste votera néanmoins en faveur de ce texte, car de la performance de nos ports maritimes dépendent la santé de notre commerce international et de notre économie et le respect de nos engagements en faveur de la transition écologique.

nos places portuaires accusent un retard par rapport à celles de nos voisins européens et sont sous-exploitées au regard de leurs potentialités, alors même que la France est la deuxième puissance maritime mondiale. Ce constat a été mis en évidence par les précédents orateurs. Il faut désormais franchir un nouveau cap. Le texte que nous examinons est la traduction législative des recommandations de la mission d'information que j'ai présidée, et dont Michel Vaspart était rapporteur. Si nous partagions beaucoup, pour ne pas dire l'essentiel, des constats et des mesures à mettre en oeuvre, nous avions quelques points de divergence, que j'ai souhaité présenter dans une proposition de loi à part, et dont certains font l'objet aujourd'hui d'amendements. Tout d'abord, nous en sommes tous d'accord, il faut que l'État définisse une stratégie nationale cohérente et ambitieuse. À cet égard, nous soutenons les mesures qui tendent à définir d'un Conseil national portuaire et logistique chargé de sa mise en oeuvre et de son suivi. C'est un besoin impérieux dans un contexte de relance économique les ports constituent en effet des lieux privilégiés de réindustrialisation, des gisements potentiels d'emplois. La création de zones franches nous apparaît opportune pour encourager l'implantation d'entreprises. le développement de nos ports ne pourra se faire sans investissements importants dans les infrastructures. Or ceux qui sont prévus par la LOM restent insuffisants. Il est indispensable de les augmenter, et nous soutenons l'ensemble des mesures financières prévues à cet effet. Une bonne gestion et une gouvernance efficace sont aussi nécessaires pour la compétitivité de nos ports : pour cela, toutes les parties prenantes doivent pouvoir participer aux décisions qui les concernent. Ainsi, les acteurs privés et les collectivités territoriales qui contribuent à leur financement et à leur fonctionnement doivent y être davantage associés. Nous saluons les mesures qui encouragent cette idée. idée. Au-delà de ces aspects, sur lesquels nous nous accordons, un point central nous sépare. Nos ports constituent un outil de souveraineté nationale pour l'approvisionnement en toutes circonstances de notre pays. La crise sanitaire l'a bien montré. En effet, les ports ont fait preuve d'une réactivité remarquable en demeurant pleinement opérationnels, assurant ainsi l'acheminement de biens essentiels, de masques et de certains produits pharmaceutiques. À l'export, ils permettent la promotion de nos filières d'excellence. Autour de cet enjeu stratégique, je dirai presque régalien, d'importants défis sont à relever dans un contexte de concurrence internationale féroce et d'urgence écologique. C'est la raison pour laquelle nous nous opposons à la possibilité ouverte de régionaliser les grands ports maritimes. L'État doit garder le contrôle de ces structures indispensables à notre indépendance et à notre économie. Pour nous, l'enjeu se situe plutôt dans la nécessaire coordination entre nos différents ports. Ils doivent jouer collectif, affronter ensemble les défis, dans une logique de complémentarité, dans le contexte du Brexit. C'est pourquoi nous attachons une importance particulière aux conseils de coordination interportuaire, dont l'article 5 améliore le fonctionnement. Nous avons souhaité que chaque façade maritime en soit systématiquement dotée. Par ailleurs, la stratégie portuaire devra inévitablement respecter nos engagements de développement durable, tant sur la question environnementale que sur la question sociale. Plus que jamais, l'économie doit se conjuguer avec les impératifs écologiques, en l'occurrence le verdissement du transport de marchandises, qui passe notamment par le fluvial. La France est le théâtre d'un grand paradoxe de ce point de vue : c'est le pays qui dispose des voies navigables les plus longues d'Europe, mais dont le taux d'utilisation est le plus faible, 80 % des acheminements reposant encore sur le routier. Pourtant, avec quatre fois moins de CO2émis que la route et sa capacité de massification importante, le fluvial est l'un des modes de transport les plus vertueux.

Or il est très réducteur de ne les envisager que sous l'angle de leur rapport avec la mer, car c'est celui avec la terre, c'est-à-dire l'hinterland, qui est défaillant et qui a freiné la constitution d'une chaîne logistique performante et écologique. Les ports sont des espaces multimodaux qu'il faut envisager dans leur prolongement vers les réseaux ferrés et fluviaux.

sera une première étape, mais il faut d'autres mesures, y compris pour la régénération de l'ensemble du réseau de voies navigables. L'établissement Voies navigables de France (VNF), tout comme SNCF Réseau, doit systématiquement être associé à la politique portuaire. Par ailleurs, pour rendre compétitif le transport fluvial face au routier, nous voulons supprimer la distorsion qu'il subit en généralisant la solution, retenue à Dunkerque, d'une mutualisation et d'une répartition uniforme des charges de manutention des conteneurs. Vous l'aurez compris, le respect de l'environnement constitue une préoccupation majeure. C'est la raison pour laquelle, malgré la nouvelle rédaction adoptée par la commission, nous demanderons la suppression de l'alinéa 3 de l'article 7, qui permettrait à un port de déroger à ses obligations de compenser toute atteinte à la biodiversité. Enfin, nos ports ne seraient rien sans les femmes et les hommes qui les font vivre, et participent indéniablement à leur essor. C'est pourquoi nous voulons que le personnel soit bien représenté au sein des conseils de surveillance. Nous veillerons également à ne pas affaiblir le modèle social auquel les salariés et les dockers sont légitimement attachés. La mise en place d'un « nouveau service minimum », alors que des règles permettent déjà de maintenir un niveau de fonctionnement suffisant de nos ports, n'est, à nos yeux, pas acceptable.

dirai que la mer peut, dans la période difficile que nous vivons, devenir une de nos plus belles opportunités, si nous défendons ensemble une politique portuaire qui préserve nos intérêts, protège nos richesses et agisse comme un moteur pour le développement des territoires,

Madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous étudions cet après-midi est le fruit d'un long travail, et d'une réflexion parlementaire qui a donné lieu à une mission d'information relative à la compétitivité internationale de nos ports. la compétitivité de nos ports, c'est aussi, bien sûr, la compétitivité de la France. Les enjeux auxquels font face nos ports maritimes sont multiples. Ils sont d'ordre économique, écologique, industriel ou encore organisationnel et géopolitique. Nos ports ont connu de nombreuses crises et, depuis 2008, ils peinent à retrouver un cap. Tout cela a été accentué par la crise du covid-19. Vous me permettrez de prendre l'exemple du port de Nantes-Saint-Nazaire, que je connais particulièrement bien puisque je suis originaire de Loire-Atlantique. Ce grand port maritime, quatrième port français, concentre tous les enjeux que j'ai déjà énumérés. (Ceser), dans un récent rapport, a fait des préconisations intéressantes pour améliorer et adapter la stratégie de Nantes-Saint-Nazaire : amorcer une diversification de l'activité, organiser la transition énergétique, notamment avec l'éolien et l'hydrogène, ou encore se coordonner avec d'autres ports de la façade Atlantique. L'une des recommandations qui a le plus attiré mon attention est celle de l'élargissement de l'hinterland. À ce titre, le fret ferroviaire ou encore les routes fluviales sont essentiels. Je salue donc la présence de représentants de VNF et de SNCF Réseau

Nous devons adapter nos ports et leur gouvernance pour les rendre plus efficaces et prospères. Comme l'a dit Édouard Philippe, alors Premier ministre, il faut des « ports entrepreneurs ». Je trouve cette expression tout à fait juste. Un plan de navigation stable à l'échelle nationale pour affronter les remous de la mondialisation est essentiel. C'est l'objectif de l'article 1 de ce texte, qui prévoit la création d'une stratégie nationale portuaire. Notre pays a une richesse maritime incroyable, l'une des plus importantes en Europe. C'est un atout pour la France et une chance pour l'Union européenne. Notre place est aux avant-postes dans la compétition internationale. Dans cette perspective, le mécanisme des zones de relance économique temporaires semble aussi pertinent. La cohérence se retrouvera également dans nos actions. Je souligne donc les avancées réalisées sur les conseils de coordination interportuaire. De la même manière, il est important d'inclure tous les acteurs en présence. J'entends par là les acteurs locaux, qu'ils viennent du monde industriel, économique ou social. Pour reprendre l'exemple du port de Nantes-Saint-Nazaire, environ 120 entreprises y sont installées, dont de très beaux fleurons français, comme Airbus ou bien encore les Chantiers de l'Atlantique. En tout, cela représente plus de 25 000 emplois, et, rien que pour le grand port maritime, plus de 80 métiers différents. Cet écosystème connaît par coeur les enjeux auxquels il fait face. Seule une association solide entre le local et le national peut rendre l'ensemble cohérent et efficient. La coordination doit également se faire entre les ports partageant une même façade. Les enjeux ne sont pas les mêmes à Marseille et à Dunkerque. En revanche, comme le montrent ses préparatifs, le Brexit nécessitera une organisation particulière, en cas de non-accord. C'est important pour notre compétitivité, notre attractivité et le respect de nos règles européennes. Enfin, je souhaite terminer par deux points.

investissant dans le verdissement des ports et du transport maritime. Deuxièmement, je veux insister sur l'article 6, qui tend à la régionalisation de la gestion des grands ports maritimes. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à connaître les discussions en cours concernant Nantes-Saint-Nazaire, mais aussi Bordeaux et La Rochelle. Je suis attaché à la décentralisation, ainsi qu'à l'inclusion des régions dans le processus décisionnel. Je crois en la subsidiarité, c'est-à-dire le principe imposant que la décision soit prise à l'échelon le plus approprié, mais je crois aussi que la stratégie nationale doit garder un poids significatif, en réponse aux enjeux de la mondialisation. La progression des nouvelles routes de la soie est mise en avant dans ce texte, mais ce n'est pas la seule stratégie. Nous devons réfléchir ensemble à une solution intermédiaire où l'État et les collectivités territoriales auraient des rôles complémentaires. La stratégie de nos ports maritimes participe de l'aménagement de notre territoire, de l'accélération de notre transition écologique et énergétique, de la garantie de notre souveraineté économique et industrielle et de l'affirmation de notre poids géopolitique dans ce monde en perpétuel mouvement. Il reste du travail, mais le Sénat sera au rendez-vous.

Si la crise sanitaire a montré la résilience de nos ports français, elle a également révélé que le modèle économique des grands ports maritimes était encore handicapé par des freins à la compétitivité. Nos portes d'entrée maritimes, qui sont bien plus que des connecteurs à l'économie mondialisée, sont devant la porte de leur propre vérité face à la concurrence de relever les nouveaux défis de ce que doit être une grande Nation maritime. Comité interministériel en 2018, Assises de la mer ... Il est temps de passer des intentions aux actes ! Malgré vos annonces à l'instant, monsieur le En préambule, je souhaite rappeler un chiffre : plus de 40 % des conteneurs à destination de la France métropolitaine transitent toujours par d'autres ports européens, principalement belges et néerlandais, et notamment Rotterdam dont a parlé Stéphane Demilly. Cette édifiante donnée motive à elle seule mon intervention sur cette proposition de loi. Ce rappel doit nous permettre de garder à l'esprit que ce texte résulte non pas d'une conjonction d'opportunités politiques, mais bien d'une volonté de pallier une politique publique défaillante. J'emploie à dessein l'adjectif « défaillant », car deux rapports dressent un panorama sans concession de la situation des ports français. Permettez-moi de citer l'un d'eux : « La performance de nos ports demeure insuffisante au regard des atouts maritimes de la France. Le rapport de juillet dernier rappelle, par ailleurs, que le projet chinois des nouvelles routes de la soie a mis en lumière le caractère stratégique des ports pour l'approvisionnement de la Nation en biens essentiels. Un autre chiffre illustre cette situation : 80 % des pré-et post-acheminements portuaires reposent encore sur le mode routier, quand 50 % du fret du port d'Hambourg est acheminé par voie ferroviaire ou fluviale. La statistique la plus éloquente est pourtant à venir : songez un instant que les six principaux ports maritimes hexagonaux représentent un total de 294 millions de tonnes de transit, le seul port de Rotterdam atteignant, de son côté, 469 millions de tonnes, et Anvers 235 millions de tonnes. Nous sommes donc face à un double défi : d'une part, nos ports manquent cruellement d'attractivité ; d'autre part, ils souffrent d'une intermodalité insuffisamment développée. Sur ce dernier point, j'ai eu l'occasion de mesurer notre retard, ayant examiné cette année en tant que rapporteur pour avis les crédits prévus dans le budget pour 2021 en faveur du transport ferroviaire, fluvial et maritime. Nous sommes particulièrement sensibles au développement de solutions de transport intermodal diversifiées, qui dépassent d'ailleurs le strict cadre portuaire. Le mode fluvial, pourtant fiable, capacitaire et capable de desservir le coeur des villes, représente seulement 2 % du transport intérieur de marchandises. La part du ferroviaire en France atteint difficilement les 9 %, alors qu'elle s'élève à 35 % en Autriche. La massification des acheminements portuaires est nécessaire à double titre : dans une optique de réduction des nuisances liées au transport de marchandises marchandises mais aussi pour renforcer la compétitivité de nos ports. En effet, comment envisager demain de gagner des parts de marché dans nos ports si, derrière, nous ne disposons pas des capacités de transport suffisantes pour absorber cette augmentation ? Comme le résume très bien la formule citée dans le rapport de la mission d'information, « à la massification maritime doit correspondre une massification terrestre ». Je salue donc les avancées prévues par la proposition de loi en la matière.

Conseil aux représentants des collectivités territoriales, des ports maritimes, de VNF, de SNCF Réseau, vont tous dans le sens du développement de solutions multimodales. De fait, cette proposition de loi suit toujours sa ligne directrice : favoriser les solutions multimodales, comme nous le constatons avec la composition et le fonctionnement des conseils de surveillance des grands ports maritimes. S'agissant du volet financier, l'augmentation de la trajectoire d'investissements de l'Afitf, fixée par la LOM, est un signal fort en faveur du fret ferroviaire et du fret fluvial. Les besoins en matière de régénération sont énormes, compte tenu des années de sous-investissement. Cette évolution pourrait d'ailleurs s'inscrire dans la stratégie nationale pour le fret ferroviaire, qui devrait, comme vous venez de nous le dire, monsieur le ministre, être présentée prochainement. Un mot, enfin, pour dire que la création d'une instance de discussion sur le surcoût de la manutention fluviale, qui serait chargée de mettre en oeuvre un plan d'optimisation à cet égard, est malheureusement devenue nécessaire. S'agissant du transport maritime, le prolongement du dispositif de suramortissement fiscal en faveur du verdissement des navires est particulièrement bienvenu, étant donnés les objectifs ambitieux, devenus impérieux en la matière, pour diminuer l'intensité carbone du transport international. Pour conclure, si ce texte est avant tout une réponse à une politique publique que nous jugeons défaillante, je m'autorise, comme mes collègues, à demander au Gouvernement, une nouvelle fois, de présenter au plus vite sa stratégie nationale portuaire, portuaire, annoncée depuis 2017. Si la France de la mer et celle de la terre ne se tournent plus le dos, le réalisme de la situation n'interdit pas d'engager formellement et rapidement plus de convergence, plus d'ambition, plus d'intermodalité, dès lors que ces objectifs sont portés et partagés politiquement aux plans national et régional. Compte tenu du contexte sanitaire, la situation des grands ports maritimes ne semble pas relever de l'urgence. Et pourtant, si nous continuons dans cette voie, nous risquons de franchir un point de non-retour. Alors, monsieur le ministre, ne repoussez pas cette proposition de loi et revenez sur votre avis initial. Aidons nos ports français à retrouver une place stratégique sur notre continent ! Ils n'ont que trop attendu. Ce texte quasi consensuel est de nature à y contribuer fortement. Monsieur le ministre, ne passez pas à côté de cette nouvelle opportunité que vous offre la Haute Assemblée.

je tiens tout d'abord à féliciter mon ancien collègue Michel Vaspart, dont l'expertise et la clairvoyance imprègnent chaque ligne de la proposition de loi que nous allons examiner. Sa passion du littoral et du domaine maritime nous manque On le sait, la France a souvent négligé sa vocation maritime, et Richelieu ne se trompait pas quand il disait que « les larmes de nos souverains [avaient] souvent eu le goût salé des mers qu'ils [avaient] ignorées pays sont pourtant extraordinaires : trois façades maritimes pour la métropole et une en outre-mer, nous donnant accès à tous les océans du globe ; un maillage portuaire composé de soixante-six ports de commerce, dont onze grands ports maritimes relevant de l'État français, à savoir sept sur le territoire métropolitain métropolitain et quatre en outre-mer- Réunion, Guadeloupe, Martinique, Guyane - ; une ZEE immense nous classant comme le plus grand territoire maritime du monde. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Le diagnostic est unanime. Ces quarante dernières années, nos ports ont pâti d'une absence de cap, d'un manque flagrant d'ambition, au plus grand bénéfice des ports étrangers. Le manque d'infrastructures, de volonté, un lobbying actif à Bruxelles de la part des ports du Benelux, le Brexit, et à présent la covid, n'ont eu de cesse de porter des coups sévères à l'émergence d'un véritable projet maritime français. Force est donc de constater aujourd'hui leur faible performance, d'une part, au regard des objectifs qui avaient présidé aux différentes réformes portuaires, et, d'autre part, en comparaison avec les autres ports européens, non seulement ceux du Nord, mais aussi ceux de la Méditerranée, rachetés de plus en plus par les Chinois. L'écart s'est déjà creusé avec nos concurrents nord-européens, mais d'autres ports étrangers, comme celui de Barcelone, semblent avoir compris que l'époque n'était plus à l'attentisme.

Venons-en aux spécificités du texte qui nous réunit. Articulée autour de cinq chapitres, cette proposition de loi vise à créer « un cadre propice à la reconquête de parts de marché pour nos ports maritimes, en particulier les grands ports maritimes relevant de l'État, têtes de pont et premières portes d'entrée du commerce extérieur français Pour y parvenir, le texte s'attache tout d'abord à refondre la gouvernance du système portuaire en introduisant plus de souplesse et une meilleure représentation de l'ensemble des acteurs concernés. C'est dans cet objectif que l'article 1 prévoit la création d'un Conseil national portuaire et logistique, chargé notamment du suivi de la stratégie nationale portuaire. Par ailleurs, et afin d'associer davantage les acteurs économiques locaux et les collectivités territoriales, la composition et le fonctionnement des conseils de surveillance des grands ports maritimes devaient être modifiés. L'article 2 s'y emploie avec pertinence. Dans le même esprit, les articles 3, 4, 5 et 6 permettraient respectivement de modifier la procédure de nomination et de révocation des directeurs généraux des grands ports maritimes, de renforcer les pouvoirs des conseils de développement, de modifier

dans le secteur des services portuaires, et notamment le remorquage, pour soutenir la diminution des coûts du passage portuaire, est une avancée importante. Le troisième défi relevé par cette proposition de loi est de tendre vers un développement portuaire en harmonie avec les questions environnementales. Nous sommes en effet convaincus que les ports maritimes jouent un rôle plus crucial que jamais dans les échanges extérieurs de l'Europe, et qu'ils sont les principaux facilitateurs multimodaux de la croissance économique de notre continent. Différentes dispositions visent donc à accompagner le verdissement du secteur portuaire par la mise à disposition d'outils incitatifs pour que les acteurs s'engagent dans la transition écologique. est ainsi de la possibilité pour les grands ports maritimes volontaires d'élaborer et de mettre en oeuvre un plan d'optimisation des coûts, ce qui permettra de favoriser le report modal et le verdissement du transport de marchandises. Je voudrais à cet égard remercier la gendarmerie maritime, qui concourt elle aussi à cette mission, en contribuant, le réseau Aquapol, à un dispositif tout à fait original en Europe visant à rendre nos ports sûrs et à en faire des facteurs déterminants d'une croissance bleue, sereine et durable. Je n'omettrai pas d'évoquer les articles 9 à 12 du chapitre III, qui visent à renforcer l'information du Parlement sur la politique portuaire. Ces articles prévoient notamment la remise de rapports du Gouvernement au Parlement sur quatre sujets. Parmi ceux-ci, la question de la progression de la stratégie la progression de la stratégie des nouvelles routes de la soie de la République populaire de Chine, me semble devoir tout particulièrement retenir notre attention. Aujourd'hui, la présence chinoise est partout visible : en Méditerranée, du Pirée à Valence, en Espagne, en passant par Marseille, Malte ou Thessalonique ; sur la côte Atlantique, à Bilbao et Nantes ; dans la Manche, au Havre ; en mer du Nord, à Dunkerque, Zeebruges, Anvers, Rotterdam, sans compter des visées sur la mer Baltique. La Chine contrôle désormais près d'un dixième des capacités portuaires européennes. Ce constat doit nous interroger plus que jamais sur notre capacité à envisager nos ports comme des éléments majeurs de notre souveraineté. Pour conclure, je dirai que tous les acteurs du milieu portuaire sont prêts à s'engager pour mettre en oeuvre les dispositifs contenus dans cette des parlementaires, mais il manque une ambition claire de l'État et de la constance pour tenir les engagements pris. Le Président Emmanuel Macron a déclaré aux Assises de la mer, le 3 décembre 2019 : « Le XXI siècle sera maritime Encore plus récemment, le gouvernement de M. Castex a réhabilité une fonction oubliée depuis la présidence de François Mitterrand, le ministère de la mer. Nous est-il permis de croire que l'heure d'une reprise en main du domaine maritime puisse sonner ? Je conclus : nous avons le devoir de redonner à la France sa grandeur d'antan, afin de laisser un merveilleux patrimoine à notre jeunesse. La parole

et qu'elle puisse franchir les portes de l'Assemblée nationale. J'espère que le débat qui va s'engager au travers de la discussion des articles permettra de mener à bien cette réforme. Encore une fois, monsieur le ministre,

par la commission, et six par Martine Filleul et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain. Ce texte est donc le fruit d'un travail élaboré en concertation avec l'ensemble des membres de la commission.

qu'ils sont chargés d'arrêter les orientations stratégiques des ports et de contrôler leur gestion. La commission a adopté un amendement du rapporteur visant à inclure un représentant de SNCF Réseau au sein des conseils de surveillance. Nous nous en félicitons, puisque nous avions proposé une telle intégration : elle permettra de favoriser le développement de l'intermodalité et de la massification des acheminements portuaires. Pour autant, afin de limiter le nombre de membres des conseils de surveillance, le rapporteur a compensé l'intégration de SNCF Réseau par la réduction du nombre des représentants du personnel des ports.

Nous considérons que ces représentants ne doivent ni être sacrifiés ni jouer un rôle de variable d'ajustement pour maintenir, à l'identique, le nombre de représentants au sein des conseils de surveillance. La représentation des salariés doit être équilibrée au regard de celle des autres membres parce qu'elle participe du bon fonctionnement du port et de la démocratie au sein des conseils de surveillance. Si le rapport de la mission d'information que j'ai présidée recommandait un resserrement des conseils de surveillance, dans un objectif d'efficacité

Cet objectif nous a permis de dégager des moyens pour relancer des autoroutes ferroviaires, dont certaines relient des ports. J'ai cité les routes de Calais-Sète, de Cherbourg-Bayonne, ou encore de Perpignan-Rungis, que nous souhaitons étendre au nord vers les ports de Dunkerque et d'Anvers, et au sud vers Barcelone.

et au développement des activités portuaires au travers d'investissements. Leur représentation au sein du conseil de surveillance, lequel arrête les orientations stratégiques du grand port maritime et exerce un contrôle permanent sur sa gestion, est donc essentielle pour éclairer les décisions contribuant à la modernisation et à la compétitivité des ports. Quel

Cet amendement vise à préserver le rôle consultatif du président du conseil de développement, qui siège au sein du conseil de surveillance. Il est vrai que la participation du président du conseil de développement

du rapport de Michel Vaspart,- adopté, je le répète, à l'unanimité en commission -a retenu un schéma proche quoique différent, en prévoyant que le président du conseil de développement soit membre de droit du conseil de surveillance.

En outre, le président du conseil de développement assure un rôle institutionnel de représentation de la place portuaire : sa présence, avec voix délibérative, est donc légitime. L'amendement conduirait également à atténuer très fortement l'évolution proposée dans le rapport de Michel Vaspart, d'où un décalage avec la position de la commission. Je demande donc le retrait de l'amendement

SNCF Réseau soient représentés au sein du conseil de surveillance. La commission a répondu en partie à notre souhait, en adoptant un amendement visant à inclure un représentant de SNCF Réseau.

grands ports maritimes. Or le fait qu'il soit représenté dans d'autres instances portuaires n'implique pas nécessairement qu'il le soit au sein du conseil de surveillance portuaire.

et de Marseille, ainsi que dans les conseils de surveillance des ports de Rouen et Paris. Il est également présent au sein des conseils de coordination interportuaire de l'axe Nord, de l'axe Seine et de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône.

oblige à choisir le président du conseil de surveillance parmi les représentants des collectivités territoriales. Sans anticiper le débat sur l'article 6 et la régionalisation

directoire. Le conseil de développement est en effet l'instance de légitimité dans la gouvernance des grands ports maritimes, du fait de sa représentativité. Nous considérons donc que les questions les plus importantes liées à la stratégie et aux investissements doivent faire l'objet d'un avis conforme en bonne et due forme. La formule adoptée par la commission, qui donne le dernier mot au directoire, tout en sommant celui-ci de se justifier, ne nous semble pas être la plus opérationnelle. Pour aller plus loin, nous estimons qu'il conviendrait de renforcer la représentativité de la commission des investissements, en y intégrant des personnalités issues des organisations syndicales représentatives du personnel. Nous proposons donc de revenir à la rédaction antérieure, qui nous semble plus respectueuse de la démocratie au sein des grands ports maritimes. Quel est l'avis de la commission

M. le ministre nous expliquera sans doute que cette rédaction initiale remettait en cause la réforme de 2008. Aussi, je vous propose de nous en tenir aux textes existants, qui ont été travaillés avec les acteurs que j'ai consultés. L'objectif est de parvenir au consensus par l'adoption d'une loi plus souple, qui permettra de renforcer le dialogue entre le directoire et le conseil de développement,

sont transmis au conseil de surveillance. Dans les faits, ces avis sont présentés par le président du conseil de développement, mais celui-ci ne peut pas participer aux délibérations du conseil de surveillance : aucun dialogue n'est donc possible autour de ses avis. L'article 2 de la proposition de loi comporte une amélioration qui nous semble essentielle, à savoir l'intégration du président du conseil de développement au sein du conseil de surveillance. Je propose, par cet amendement, d'apporter une précision supplémentaire, afin de favoriser un dialogue fluide entre les instances. L'amendement vise à ce que le président du conseil de développement présente les avis rendus par ce dernier devant le conseil de surveillance, et assiste aux délibérations portant sur ces avis. Quel

pour les régions qui en feraient la demande, d'un transfert en pleine propriété de grands ports maritimes. Je considère que la rédaction de cet article

demeurent une compétence de l'État. Les ports sont des maillons stratégiques indispensables à la performance et à la résilience des chaînes logistiques. À l'export, ils permettent la promotion de nos filières d'excellence. Ils sont un outil de souveraineté nationale pour l'approvisionnement en toutes circonstances de notre pays, comme l'a démontré la crise sanitaire. Les infrastructures portuaires ont en effet permis d'assurer la continuité des approvisionnements en produits essentiels à la vie de notre pays, qu'il s'agisse des produits agroalimentaires ou du matériel médical. Par ailleurs, en admettant que les collectivités soient à même de gérer ces grands ports, qui nous dit qu'elles ne seront pas tentées, voire contraintes, de céder ces actifs, et pourquoi pas à des pays comme la Chine qui mène une politique active d'acquisitions partout et dans de nombreux domaines ? Qu'est-ce qui nous protège de ce type d'éventualité ? C'est alors une part de notre souveraineté nationale que nous abandonnerions

ne s'y sont pas intéressés et d'autres y étaient totalement opposés, à l'exception du grand port de Bordeaux et de la région qui pourraient être intéressés. La décentralisation risque d'être particulièrement pénalisante si les collectivités territoriales ne disposent pas de moyens importants pour assumer cette nouvelle compétence. Troisième raison, nous redoutons que la régionalisation ne se traduise

Un tel transfert aux collectivités territoriales de la gestion des grands ports maritimes n'est pas opportun puisque l'importance et le rayon d'action de ces ports dépassent largement les enjeux de la région où ils sont À titre d'exemple, Dunkerque a vocation à desservir les Hauts-de-France, l'Île-de-France mais aussi le Grand Est. Haropa a une aire d'influence sur toute la moitié nord de la France et une partie de la façade atlantique, potentiellement jusqu'en Nouvelle-Aquitaine.

En effet, il est à craindre que ce transfert de compétence portuaire à l'échelle régionale mène non seulement à une situation d'immobilisme et à une absence de formulation de stratégie de développement national, mais aussi à un manque de coordination des investissements entre des entités appartenant à des aires administratives distinctes.

je ne développerai pas la situation de tension que vivent ces collectivités territoriales. Voilà au moins quatre raisons qui nous conduisent à demander la suppression de cet article.

plus que d'un article de droit. Compte tenu du fait que les ports nationaux relèvent d'une politique nationale, que celle-ci n'a pas l'ampleur qu'il faudrait lui donner, je me demande si nous ne devrions pas nous orienter plutôt vers l'exigence que le Gouvernement s'implique davantage dans le développement de cette activité portuaire. Quand j'entends dire que l'activité du port du Havre a diminué de 28 % l'année dernière, je m'inquiète pour l'avenir de nos ports nationaux. Je ne suis pas sûr que le démantèlement d'une politique nationale n'ayant pas produit les effets que l'on en attend soit véritablement la solution pour redonner

par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrage. Ces mesures de compensation ne peuvent pas se substituer aux mesures d'évitement ou de réduction. Si les atteintes liées au projet ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, celui-ci n'est pas autorisé en l'état. Les mesures doivent alors être mises en oeuvre en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci, afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne.

2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a fixées en matière de compensation des atteintes à la biodiversité, et qui sont codifiées à l'article L. 163-1 du code de l'environnement. En commission, le rapporteur a proposé un amendement, qui devrait permettre de répondre à nos inquiétudes, mais à ce stade, nous ne sommes toujours pas convaincus par la rédaction actuelle de l'article 7, qui vise à mieux concilier les mesures de compensation prévues par le droit de l'environnement et les projets stratégiques des ports. En quoi le fait de prévoir une prise en compte plutôt qu'une compatibilité permettrait-il de limiter les éventuelles dérogations qui pourraient être apportées aux mesures de compensation prévues par le droit de l'environnement ? Le fait de limiter ces dérogations ne les supprime pas pour autant. Sauf démonstration contraire, nous continuons de penser que les alinéas 2 et 3 pourraient servir à contourner l'obligation de compensation des atteintes à la biodiversité.

à la mise en oeuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité prévues à l'article L.163-1 du code de l'environnement. Les questions environnementales sont décisives, en particulier la préservation de la biodiversité dans l'espace portuaire. L'article L.163-1 du code de l'environnement prévoit que la mise en oeuvre des mesures de compensation doit être réalisée en priorité sur le site endommagé ou, en tout état de cause, à proximité de celui-ci, afin de garantir ses fonctionnalités de manière pérenne. Pour Michel Vaspart, rapporteur de la mission qui a présidé à la rédaction de la présente proposition de loi, il convient d'appliquer le principe de proximité avec une approche fonctionnelle : « La compensation écologique pourrait notamment être utilisée pour développer des ceintures vertes autour des ports, renforçant leur intégration dans leur environnement et la préservation de ce dernier. » Il est donc possible de concilier développement portuaire et préservation de l'environnement, sans pour autant déroger à la mise en oeuvre des mesures de compensation dans le cadre du futur développement des ports. C'est pourquoi cet amendement vise à s'assurer que les mesures de compensation prévues par le droit de l'environnement et les projets stratégiques des ports sont en cohérence, tout en conservant un haut niveau de protection de l'environnement. La référence à une dérogation n'apparaît donc pas nécessaire et crée une ambiguïté inutile.

objectif est de trouver un équilibre entre la nécessité de conserver un haut niveau de protection de l'environnement, d'une part, et celle de créer les conditions du développement futur des ports, d'autre part. La mise en oeuvre de mesures de compensation des atteintes à la biodiversité qui peuvent résulter des travaux engagés par les ports

et que les dérogations prévues sont limitées, puisqu'il s'agit d'une simple prise en compte du projet du port, et non d'une exigence de compatibilité lors de la mise en oeuvre des mesures de compensation. Dans certains

velléités de certains d'établir un véritable service minimum pour le remorquage portuaire, avec une extension des pouvoirs de réquisition du président du directoire grand port maritime, ont été écartées. Elles n'étaient pas sans rappeler les différentes tentatives d'imposer des exigences supplémentaires en matière de garanties de service minimum, qui remettent en cause, selon nous, le droit de grève. Je pense notamment à la proposition de loi de Bruno Retailleau visant à réquisitionner du personnel, y compris gréviste, pour assurer un service minimum dans les transports publics du quotidien, de loi de M. Guerriau portant obligation de déclaration d'un préavis de grève des contrôleurs aériens, ou encore à la tentative, lors de l'examen de la LOM, de porter de quarante-huit à soixante-douze heures le délai de la déclaration individuelle de grève dans les transports publics terrestres. Comme dans les cas cités précédemment, nous estimons que les grèves témoignent avant tout de l'absence de dialogue social ou d'une mauvaise qualité de celui-ci. Selon nous, le renforcement des exigences en matière de service minimum risque d'être contre-productif, voire d'envenimer les conflits. Même dans une version « soft », comme celle qui est proposée dans cet article, nous demeurons dubitatifs quant à l'efficacité de telles mesures. Tout d'abord, il existe un règlement européen de 2017 qui donne la possibilité aux autorités portuaires de fixer les exigences minimales de service public. Or, par définition, les règlements européens sont d'application directe. Ensuite, la création d'un service minimum pour le remorquage serait contraire au droit actuel, le Gouvernement ayant souligné dans sa réponse aux questions posées par le rapporteur que les agréments pouvaient imposer la continuité du service, permettant ainsi de garantir la disponibilité du service portuaire pour l'ensemble des utilisateurs sans interruption. Le renforcement des exigences de service minimum pour une activité comme le remorquage, qui ne constitue pas un véritable service public, est périlleux. Pour toutes ces raisons, nous nous opposons à ces dispositions qui visent à renforcer

comme un simple dispositif permettant de garantir un niveau de qualité et de disponibilité des services portuaires, en particulier du remorquage, et de favoriser une dynamique concurrentielle. En réalité, derrière les mots se cache un objectif, celui d'aller vers la mise en oeuvre d'un service minimum portuaire,

La compétitivité des ports ne pourra pas se renforcer au détriment des droits des salariés. Jeter le discrédit sur le coût du travail est une opération fallacieuse. Doit-on rappeler qu'un travailleur portuaire a une espérance de vie de sept ans inférieure à la moyenne Par ailleurs, en s'adossant au règlement européen, et en appelant à une convention entre les entreprises de remorquage et l'autorité compétente de l'État pour déterminer l'organisation du dialogue social et les modalités de prévention des conflits, vous laissez croire que le règlement européen permet l'instauration d'un tel service minimum. Il n'en est rien, puisque l'article 7 de ce règlement dispose que les actions sociales collectives menées conformément au droit national ne sont pas considérées comme des cas de perturbations des services portuaires. Le fondement juridique d'une telle limitation n'est donc pas avéré au niveau européen. Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article, qui n'est pas propice à l'amélioration du dialogue social dans les grands ports maritimes. Quel

conduiraient à imposer un service minimum. Elles me paraissent en outre poser deux types de difficultés : d'une part, des difficultés juridiques, car cela reviendrait à réquisitionner des personnels d'entreprises privées qui ne sont pas en charge de l'exécution d'un service public, ce qui porterait vraisemblablement une atteinte disproportionnée au droit de grève et à la liberté d'entreprendre ; d'autre part, des difficultés sociales,

Afin de réellement favoriser et d'engager le report modal vers le transport ferroviaire et le transport fluvial, nous considérons qu'il convient de réguler les pratiques. les pratiques. Cet amendement vise à aller au-delà de la simple possibilité de prévoir, dans les conventions de terminal, une part dégressive du montant de la redevance due en fonction de la performance environnementale de la chaîne de transport. Il prévoit ainsi l'obligation d'introduire des clauses financières liées à des critères environnementaux, afin que des objectifs contractualisés de part modale, conjugués à un signal prix tenant compte des externalités, soient mis en place par les ports.

cette mesure. Cet amendement tend également à supprimer la modulation de la redevance en fonction du trafic pour ne garder que la modulation en fonction de la performance environnementale de la chaîne de transport, la première mesure pouvant entrer en contradiction avec la seconde, et réciproquement. Il s'agit ainsi de n'encourager que les pratiques vertueuses et respectueuses de l'environnement. Enfin, nous proposons de fixer un objectif minimum de recours aux modes massifiés- d'au moins 20 % -pour les grands ports maritimes disposant d'un accès ferroviaire ou fluvial.

Depuis la réforme portuaire, les tarifs facturés par les entreprises de manutention aux opérateurs fluviaux augmentent considérablement. Or l'opérateur fluvial, qui ne maîtrise pas l'opération logistique de bout en bout, n'a ni le choix du terminal ni celui de l'opérateur de manutention, sur lequel il n'a aucun moyen de pression commercial. S'agissant du transport routier et ferroviaire, la règle en vigueur est que l'ensemble des coûts de la manutention portuaire est facturé au donneur d'ordre. Cette situation

Ces dernières années, nombreuses ont été les initiatives pour remédier à cet état de fait, en particulier dans le grand port maritime de Dunkerque, et ce à partir de septembre 2015. Le bilan de l'expérimentation réalisée a conclu à un succès indéniable de cette opération, fondée sur la prise en charge par les armateurs maritimes de ce coût, et non sur une mutualisation de tous les modes de transport. Il est attesté par la progression significative des trafics, qui ont été multipliés par deux en moins d'un an, et par l'adhésion de la totalité des acteurs de la place au dispositif. Ces nouvelles modalités de facturation de la manutention sont la règle au grand port maritime de Dunkerque depuis le 1 janvier 2017. Or les rapports parlementaires sur l'attractivité des ports français, remis au secrétaire d'État en juillet 2016, fixent tous comme priorité le rééquilibrage des coûts de manutention des conteneurs pour le transport fluvial. Ils confirment qu'ils sont un déterminant important de la compétitivité du transport fluvial.

évoquer les grands échanges organisés par l'Europe. Je pense en particulier au corridor Atlantique que l'Europe veut mettre en place, c'est-à-dire un ensemble de ports qui permettraient d'assurer un acheminement correct des marchandises. les candidats à ce corridor, on trouve notamment les ports de Brest et de Roscoff, qui se situent à la pointe de la Bretagne et qui voient passer la plupart des porte-conteneurs

effectif qui assure une intermodalité. Cela suppose notamment que le système européen de signalisation soit mis en oeuvre un peu partout.

Je tiens à renouveler mes remerciements aux auteurs de cette proposition de loi, à saluer l'engagement de chacune et chacun d'entre vous, mes chers collègues, et la qualité de nos échanges. Je n'exprimerai qu'un tout petit regret. Quel dommage que le Sénat, représentant des collectivités territoriales, ait raté l'occasion de prévoir que la présidence du conseil de surveillance revienne à un membre du collège des élus locaux ! C'était pourtant

et sénatoriales partielles, et un projet de loi relatif aux délais d'organisation des élections municipales partielles et des élections des membres des commissions syndicales. Une fois encore, Il a été décidé que ces deux textes feraient l'objet d'une discussion générale commune.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

Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, madame la rapporteure, mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, je suis heureuse d'être parmi vous ce soir pour vous présenter ces projets de loi, qui concernent l'organisation de notre vie démocratique dans un contexte sanitaire inédit. Le rythme de circulation du virus responsable de la covid-19 s'est, comme vous le savez, de nouveau accéléré en octobre et les circonstances sanitaires peuvent compromettre momentanément l'organisation d'élections sur le territoire national- plus que le scrutin encore, la campagne qui les précède. Or, dans cette période sans équivalent, se créent des situations de vacances de siège dans les assemblées élues. Certaines sont déjà constatées ; d'autres sont à prévoir. Ces vacances de siège ont déclenché ou sont susceptibles de déclencher l'organisation d'élections partielles. Ainsi, une élection législative partielle devait avoir lieu prochainement dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais. Une autre est à prévoir dans la quinzième circonscription de Paris. À ce jour, environ 160 élections municipales partielles doivent aussi être organisées. Or le code électoral fixe un délai de trois mois pour organiser ces élections partielles. Un tel délai est apparu impossible à respecter dans le contexte sanitaire actuel, lorsque l'organisation d'une élection partielle implique, par exemple, le déplacement d'un grand nombre d'électeurs dans une zone de forte circulation du virus. C'est pourquoi le Gouvernement soumet à votre assemblée les projets de loi organique et ordinaire que nous allons examiner ce soir. Plus précisément, le projet de loi organique tend à permettre, si la situation sanitaire l'exige, une convocation des élections législatives et sénatoriales partielles au-delà du délai de trois mois prévu par les dispositions de droit commun. Le projet de loi ordinaire procède de même s'agissant des élections municipales partielles.

Ce n'est donc pas un report absolu et général ; la situation doit être appréciée en tenant compte de la situation locale. La commission des lois de votre assemblée a souhaité introduire des garde-fous supplémentaires pour encadrer cette possibilité de report des élections partielles.

partielle dont le générateur intervient le 15 février pourrait être organisée jusqu'au 13 juin, alors qu'une élection partielle déclenchée le 17 février, c'est-à-dire deux jours plus tard, devrait obligatoirement se tenir avant le 17 mai.

Si la logique de subsidiarité sous-tendant cette disposition se conçoit aisément, sa mise en oeuvre pourrait, elle, se révéler plus complexe, avec un risque de divergence dans les méthodes d'objectivation de la situation sanitaire.

L'un est organique et concerne les élections législatives et sénatoriales partielles ; l'autre porte sur les élections municipales et métropolitaines et, à titre subsidiaire, sur les commissions syndicales dans les sections de commune. Ces élections partielles auraient lieu

les projets de loi doivent être promulgués avant la fin du mois de décembre, notamment pour acter le report des élections législatives partielles dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais. Le Sénat est appelé à délibérer seulement quatre jours après l'Assemblée nationale, alors que le Gouvernement a annoncé le dépôt d'un autre texte pour reporter les élections régionales et départementales prévues en mars 2021. Dans ses projets de loi initiaux, le Gouvernement s'est même abstenu d'étendre certaines dispositions aux collectivités d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie pour éviter de consulter les assemblées territoriales. Cette extension a été opérée par les députés, ce qui semble respecter la jurisprudence du Conseil constitutionnel mais pas l'esprit de nos institutions. Je souhaite dire ici que le Sénat ne cautionne pas cette manière de procéder, qui laisse à l'écart les assemblées d'outre-mer. Les conditions d'un débat serein et éclairé sont donc loin d'être réunies. réunies. Face aux incertitudes liées à l'épidémie de covid-19, nous pouvons toutefois admettre la nécessité du report des élections partielles. Le code électoral prévoit, en effet, un délai de trois mois pour organiser ces scrutins, ce qui conduirait à les organiser pendant la seconde vague de l'épidémie. Deux sièges sont vacants à l'Assemblée nationale. Dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais, je l'ai dit, l'élection aurait dû se dérouler avant le 27 décembre 2020. Dans la quinzième circonscription de Paris, l'élection doit se dérouler avant le 20 février 2021. À l'échelle locale, des élections municipales partielles doivent être organisées dans 161 communes au moins. Le nombre d'élections pendantes augmente toutefois au fil des semaines, en fonction des décès, des démissions de conseillers municipaux, mais également du calendrier des contentieux. De nouvelles annulations sont d'ailleurs à prévoir dans les prochaines semaines, le juge électoral n'ayant pas encore « purgé » l'ensemble des recours qui lui ont été soumis. Ainsi, en raison de la crise sanitaire, et dérogeant au droit commun, le Gouvernement souhaite allonger temporairement le délai d'organisation des scrutins partiels pour : les élections municipales, les élections dans les arrondissements de Paris, Lyon et Marseille et les élections à la métropole de Lyon ; l'élection des membres des commissions syndicales dans les sections de commune ; les élections législatives et sénatoriales. l'initiative du Gouvernement, l'Assemblée nationale a ajouté à ce périmètre les élections territoriales partielles des collectivités d'outre-mer, ainsi que les élections partielles pour les assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie. Ces élections partielles seraient organisées dès que la situation sanitaire le permettra, et au plus tard le 13 juin 2021. Il s'agit bien d'une date butoir : l'autorité administrative devra organiser les élections partielles le plus tôt possible, notamment dans les départements les moins touchés par le virus. Le Gouvernement s'y est engagé dans son étude d'impact. Le calendrier électoral pourrait donc varier d'une circonscription à l'autre, en fonction des circonstances locales. Sur le terrain, l'autorité administrative a d'ores et déjà annulé plusieurs élections plusieurs élections partielles prévues d'ici à la fin de l'année 2020, en l'absence de texte, mais en s'appuyant sur la théorie des circonstances exceptionnelles. Elle a ainsi dérogé au délai d'organisation de trois mois pour l'élection législative partielle dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais et pour 26 élections municipales partielles. En revanche, plus ponctuellement, certains sous-préfets ont continué d'organiser des élections partielles pendant le confinement, notamment dans les départements de la Marne et du Tarn-et-Garonne. Sur le plan juridique, je rappelle que nous avons déjà reporté plusieurs scrutins en raison de la crise sanitaire, dont le second tour des élections municipales, les élections consulaires des Français de l'étranger et l'élection de six sénateurs représentant les Français établis hors de France. De même, certaines élections partielles ont été « gelées » pendant le premier confinement. relative à la loi d'urgence du 23 mars 2020, le Conseil constitutionnel a confirmé que l'impératif sanitaire pouvait justifier un report des élections et, donc, des aménagements au principe de périodicité raisonnable du scrutin. Toutefois, si la situation sanitaire justifie le report des élections partielles, le cas échéant jusqu'au 13 juin 2021, ce n'est pas sans conséquences concrètes sur le fonctionnement des conseils municipaux. Deux situations d'inégale gravité peuvent ainsi se présenter. Dans certaines communes de moins de 1 000 habitants, des élections partielles « complémentaires » sont nécessaires pour compléter le conseil municipal. C'est le cas de 101 communes sur les 161 soumises à élections partielles. Dans l'attente, le conseil municipal continue de fonctionner et dispose de l'ensemble de ses compétences. En cas de décès du maire, l'intérim est assuré par l'un de ses adjoints. Dans les 60 communes restantes, une délégation spéciale a été mise en place, notamment lorsque l'élection a été définitivement annulée. Or les pouvoirs des délégations spéciales sont limités à la gestion des affaires courantes, ce qui peut créer des complications pour apporter une réponse aux conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. En raison du report des élections partielles, les délégations spéciales seraient donc mises en place pour une période qui pourrait dépasser trois mois. Sur le terrain, cette « paralysie » de l'administration municipale pourrait soulever des difficultés au regard du principe de libre administration des collectivités territoriales. Conscient de cette difficulté, le Conseil d'État a invité le Gouvernement à prendre en considération les conséquences du report des élections partielles sur le fonctionnement des conseils municipaux ; seul un motif sanitaire « impérieux » peut justifier le report des scrutins dans les communes où une délégation spéciale a été installée. Il faudra donc y veiller pour chacune des communes concernées. De jurisprudence constante, le report d'une élection doit respecter deux conditions : d'une part, le législateur doit définir avec suffisamment de précision le calendrier électoral et, ainsi, éviter tout risque d'incompétence négative ; d'autre part, le report d'une élection doit être exceptionnel, transitoire, mais aussi proportionné à l'objectif d'intérêt général visé. Aussi, la commission des lois a souhaité introduire plusieurs garde-fous, comme vient de l'expliquer Mme la ministre, pour s'assurer que l'administration convoque ces scrutins dès que la situation sanitaire le permettra et, si cela est possible sur le plan sanitaire, avant le 13 juin 2021. En premier lieu, nous avons proposé de revenir plus rapidement au régime de droit commun : la possibilité de reporter les élections partielles s'appliquerait aux vacances de siège survenues avant le 16 février 2021, et non le 13 mars, en cohérence avec la date de sortie de l'état d'urgence sanitaire. Les vacances de siège survenues entre le 17 février et le 13 mars 2021 seraient donc traitées dans les conditions prévues par le code électoral, avec l'organisation d'une élection partielle dans un délai de trois mois. En deuxième lieu, nous souhaitons remplacer les « recommandations générales » du comité de scientifiques, qui ne permettraient pas d'apprécier la situation sanitaire spécifique à chaque circonscription, par des rapports circonstanciés des ARS, présentés

En dernier lieu, nous souhaitons introduire une voie de recours spécifique pour que les électeurs puissent contester le refus par une autorité administrative de convoquer des élections partielles, alors que la situation sanitaire le permettrait. L'autorité administrative disposerait d'un délai de quinze jours pour répondre à la requête de l'électeur, son silence valant rejet. L'électeur pourrait ensuite saisir le juge des référés, qui se prononcerait en quarante-huit heures sur la possibilité, ou non, d'organiser les élections partielles au regard de la situation sanitaire. Enfin, la commission des lois a ajouté deux dispositifs pour sécuriser les conditions d'organisation de ces élections partielles, en s'inspirant du dispositif mis en oeuvre pour le second tour des élections municipales du 28 juin 2020. Premièrement, l'État prendrait en charge les équipements de protection à destination des électeurs et des membres des bureaux de vote, et s'occuperait de fournir les communes. Deuxièmement, outre la double procuration introduite par l'Assemblée nationale, le recours aux procurations serait facilité pour les personnes vulnérables, qui pourraient en établir une depuis leur domicile, sans justificatif, notamment sur simple appel téléphonique ou, le cas échéant, par voie électronique. Ce dispositif ne s'appliquerait pas aux élections sénatoriales partielles, en raison de la spécificité de ce scrutin et du recours plus limité aux procurations. Je vous invite, mes chers collègues, à adopter le projet de loi organique et le projet de loi ainsi modifiés. Madame la ministre, mes

En accord avec la commission des lois et le Gouvernement, nous pourrions, à l'issue de la discussion générale, suspendre brièvement la séance pour permettre à la commission de les examiner et reprendre immédiatement nos travaux,

-pour fixer la date d'une élection partielle après la vacance d'une institution ou d'un siège. Cette extension vise à minimiser les risques sanitaires pour

n'entraînera pas de contacts interpersonnels très intenses ou démultipliés, le délai normal de trois mois pourra sans doute être retenu

d'annonces de déferlements contentieux ayant suivi les élections municipales, le nombre d'annulations qui vont donner lieu à des élections partielles est tout à fait conforme aux « récoltes » antérieures. Comme chaque fois que j'en ai l'occasion, je veux rendre hommage au sérieux, au professionnalisme et à la rigueur juridique avec lesquels les tribunaux administratifs ont accompli leur office pour ces différentes élections. Donc nous disposerons de cette marge d'adaptation,

Ainsi, en choisissant la date du 16 février pour servir de point de départ au délai maximal de trois mois, nous ne faisons pas grande différence. Il me semble donc que nous allons pouvoir nous rassembler autour de cette mesure et, après

La parole est à M. Jean-Yves Roux. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le projet de loi organique que nous examinons aujourd'hui prévoit, dans un article unique, la possibilité de reporter les élections partielles pour les députés et les sénateurs au-delà du délai de trois mois après la constatation de la vacance de leur siège. L'organisation du scrutin interviendrait alors en fonction de l'état sanitaire de la France et, au plus tard, le dimanche 13 juin 2021. Le projet de loi ordinaire prévoit, pour sa part, les mêmes dispositions pour les élections partielles relatives à un siège de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement, l'article 2 modifiant quant à lui les élections des membres des commissions syndicales. Le Parlement ayant autorisé la prolongation de l'état d'urgence au 16 février 2021, il paraît effectivement cohérent que nous puissions, dans ce contexte précis, adapter en conséquence les dates de ces prochaines échéances électorales. Les Français ne comprendraient pas que nous leur demandions des efforts et que nous n'agissions pas de même pour faire vivre notre démocratie. Des circonscriptions, certes minoritaires, ne peuvent rester sans député indéfiniment. Des territoires ne peuvent rester sans représentants.

Ce qui fonde notre démocratie représentative, ce n'est pas seulement l'organisation optimale et sincère des scrutins ; c'est la possibilité d'organiser des campagnes électorales permettant à chacun de poser les enjeux des scrutins, comme les compétences territoriales. Nous sommes à ce titre soucieux que l'État propose, en appui, des campagnes institutionnelles de qualité, clairement identifiées, adaptées aux nouveaux moyens de communication comme aux circonstances sanitaires. Le rapport confié à Jean-Louis Debré, rendu public le 13 novembre, établit par ailleurs des recommandations de bon sens, que nous jugeons nécessaire de prendre en compte pour tous les scrutins électoraux À des fins d'organisation mais aussi de lisibilité démocratique, nous souhaitons, dans la mesure du possible, que la totalité de l'échéancier électoral soit connue le plus vite possible. Nous savons que nous sommes dépendants de l'évolution sanitaire et des campagnes vaccinales du premier semestre 2021, mais les Français ont besoin de perspectives et d'un cadre démocratique pour se projeter. Nos élus et notre administration territoriale doivent pouvoir s'organiser en amont pour l'établissement et la réactualisation des listes électorales. Nos maires et leurs équipes doivent pouvoir informer suffisamment en avance des nouvelles modalités de vote, notamment des votes par procuration, et assurer ainsi une parfaite sincérité du scrutin. Concernant les campagnes électorales, nous sommes effectivement attentifs à la proposition n° 4 du rapport de Jean-Louis Debré, mentionnant la nécessité d'« aménager les conséquences du report des scrutins sur la conduite des campagnes électorales ». Nous souhaitons aussi des éclaircissements sur les règles applicables au cumul en cas de multiples candidatures le même jour. Le RDSE est par ailleurs très vigilant à ce que la dignité des personnes soit pleinement préservée, malgré le caractère exceptionnel de l'organisation de ces scrutins. La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice avait posé les bases d'une plus grande indépendance du vote des personnes plus fragiles. Dans un contexte sanitaire où il pourrait être encore difficile d'organiser des campagnes électorales pleinement égalitaires dans les établissements accueillant des personnes âgées, nous souhaitons que la visite d'officiers de police judiciaire, dans le respect des gestes barrières, puisse être facilitée pour accompagner ces personnes dans leur choix. Je terminerai par la question du vote par correspondance. Les travaux de la commission des lois se poursuivent avec sérénité et sérieux. Je ne doute pas que le Gouvernement aura à coeur de prendre en compte les propositions et remarques de la Haute Assemblée pour avancer sur cette question. Le RDSE votera ces projets de loi.

viennent s'ajouter à la liste des dispositions que nous votons, depuis maintenant plusieurs mois, pour contrecarrer les conséquences de l'épidémie de covid-19. Nous le savons, cette crise met sous cloche la vie sociale, en général, et malheureusement une de ses composantes essentielles, la démocratie.

scrutins, d'égalité entre les candidats, de bonne information des électeurs ou encore des impératifs de transparence. Pourquoi le Gouvernement a-t-il attendu pour nous transmettre ces textes ? Nous nous retrouvons à devoir les examiner de manière précipitée en commission, ce matin, et en séance, cet après-midi. Cela illustre le peu de respect de l'exécutif envers le Parlement, qui devrait acter machinalement ses volontés. Nous saluons d'autant plus le travail de la commission des lois.

utilement, que l'État devait se porter garant des bonnes conditions matérielles d'organisation du scrutin. Les élections ne sont pas une formalité. Ce sujet à l'apparence technique ne peut donc pas être pris à la légère et glisser ainsi dans notre ordre du jour. Cette précipitation semble liée à un cas particulier, celui de l'élection partielle dans la sixième circonscription du Pas-de-Calais. Au-delà de la forme, le fond de ce texte soulève certains problèmes.

13 juin prochain semble d'autant plus à contre-courant qu'on nous les présente au moment même où l'on déconfine le pays. La démocratie, aussi, doit être déconfinée Le Gouvernement le doit aux représentants des forces politiques, aux élus locaux et aux citoyens. Nous ne sommes pas dans la même situation que pour les élections municipales. Les élections partielles sont circonscrites

que la tenue des élections est un sujet éminemment politique : ce n'est pas une simple case à cocher, un simple report à décider ! Cela implique des campagnes bousculées, des façons d'informer à réinventer, des moyens à donner aux candidats et aux organisateurs pour assurer, au-delà du de ces élections, la visibilité et la consistance républicaine qui y est attachée. Les effets de la crise ne doivent plus être des surprises quotidiennes ; le Gouvernement aurait dû prendre ses responsabilités pour mieux anticiper les échéances électorales. C'est un constat global depuis les municipales puisque, s'agissant des élections départementales et régionales, nous sommes toujours dans l'attente du projet de loi qui devrait les reporter à juin prochain, avec un risque non négligeable de concomitance avec des élections partielles. Ces élections structurent la vie citoyenne de notre pays ; certaines attentes des élus et des citoyens ne sauraient être bâclées. S'il est nécessaire d'apporter des réponses aux situations locales en suspens, nous souhaitons que le Gouvernement sorte d'une stratégie de l'improvisation constante.

encore, cet examen intervient dans un contexte très particulier, celui de la crise sanitaire que connaît notre pays. Cette crise a eu indéniablement des conséquences sur la vie démocratique. En effet, en raison de la circulation active du virus sur tout le territoire national, dès l'arrivée de la première vague, le législateur a dû adapter à plusieurs reprises le calendrier électoral tout en suivant les recommandations du conseil scientifique covid-19. Il a ainsi été amené à reporter le second tour des élections municipales en juin dernier, les élections consulaires, le renouvellement de six de nos collègues sénateurs représentant les Français de l'étranger, ainsi que les élections départementales partielles qui auraient pu intervenir pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire. Aujourd'hui encore, la circulation du virus est très active. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il nous est donc nécessaire de statuer sur le report des élections partielles. Rappelons que celles-ci interviendraient en cas de vacance d'un siège de député, de sénateur, de conseiller municipal ou encore de membre d'une organisation syndicale. Tout au long de notre discussion, il sera important de garder à l'esprit que nous devons concilier deux impératifs fondamentaux : la continuité de la vie démocratique, d'une part, et la préservation de la santé publique de nos concitoyens, d'autre part.

ce même report étant autorisé par le projet de loi ordinaire pour les élections municipales partielles. Quoi qu'il en soit, ces scrutins devront se tenir au plus tard le 13 juin 2021. Adoptés en fin de semaine dernière par l'Assemblée nationale, ces deux textes n'ont quasiment pas été modifiés par nos collègues députés, à l'exception de l'ajout d'une disposition prévoyant, sur le modèle de ce que nous avions retenu pour les dernières élections municipales, qu'un électeur pourra disposer de deux procurations. Je tiens à remercier notre collègue Catherine Di Folco, rapporteur de la commission des lois, de son travail, de son rapport et de sa volonté de parvenir à un consensus afin que notre démocratie, malgré la progression de l'épidémie, continue de s'exercer de la manière la plus normale qui soit. La commission des lois de notre Haute Assemblée, même si elle ne remet pas en cause ces reports en raison du contexte épidémiologique, a souhaité apporter quelques aménagements. Nombre de nos concitoyens résidant dans des communes où des élections doivent ou devaient se tenir se retrouveront administrés par des délégations spéciales,

Cependant, mes chers collègues, vous constaterez que cette situation est peu satisfaisante d'un point de vue démocratique. C'est pourquoi notre commission a retravaillé le texte afin d'éviter au maximum que cette situation ne perdure dans le temps, en incitant à organiser les partielles dès que la situation sanitaire le permettra.

cette proposition émanât du Sénat. Il s'agit d'inscrire dans la loi que les ARS, dans les cas où des élections partielles devaient se tenir dans une commune de leur région, rendent leur avis sur la possibilité ou non d'organiser ce scrutin. Dans la mesure où, depuis le début de la pandémie, ces agences publient quotidiennement les chiffres de l'état sanitaire de leur territoire, il nous a semblé souhaitable de procéder à ces modifications. Enfin, notre attention s'est portée sur les recours que pourrait intenter tout citoyen à défaut d'organisation d'un scrutin par le préfet, alors que la situation sanitaire le permettrait. L'autorité administrative disposerait de quinze jours pour répondre à la requête de l'électeur, son silence valant rejet. Il appartiendrait ensuite au juge des référés de se prononcer sous quarante-huit heures sur la possibilité ou non d'organiser les élections. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, ces modifications tendent à ce que les différentes élections qui devraient se tenir l'an prochain soient espacées, autant que faire se peut, dans le temps. En effet, les élections partielles pourront, aux termes des textes que nous examinons aujourd'hui, être reportées au plus tard au 13 juin 2021, mois durant lequel devraient se tenir,

Il en est de même sur le plan démocratique, avec le report du second tour des élections municipales et l'installation tardive des équipes communales et communautaires. Aujourd'hui, le Gouvernement sollicite du Parlement, dans l'urgence, de reporter l'élection législative partielle de la sixième circonscription du Pas-de-Calais, ainsi que celle de la quinzième circonscription de Paris. Ce projet de loi organique, qui prend en considération ces deux vacances de poste et celles qui pourraient advenir tant à l'Assemblée nationale arrive tardivement, alors que le second confinement a été décidé le 29 octobre, que l'état d'urgence sanitaire a été reconduit le 14 novembre et que l'élection législative partielle du Pas-de-Calais devait avoir lieu les 13 et 20 décembre prochain. De ce point de vue, madame la ministre, il est regrettable et déplorable que les candidats, alors qu'ils étaient en campagne et qu'ils avaient préparé leurs documents, n'aient été prévenus par un mail de la préfecture que le 25 novembre de l'annulation des commissions de propagande des 30 novembre et 16 décembre,

Tout siège de député qui deviendrait vacant après le 1 mai le resterait jusqu'au prochain renouvellement, de même que tout siège qui ne ferait pas l'objet d'un renouvellement avant cette date si la situation sanitaire ne le permettait pas. Un report aussi lointain ne nous paraît ni souhaitable ni acceptable. D'une part, la situation sanitaire s'améliorant quelque peu, le Président de la République a annoncé un calendrier de déconfinement progressif ; d'autre part, l'état d'urgence sanitaire prend fin le 16 février prochain.

Avons-nous la certitude pour autant que, à cette période, la situation sanitaire sera maîtrisée ? Non. Mais il n'en demeure pas moins que, s'agissant de la sixième circonscription du Pas-de-Calais, dont le scrutin se tiendrait le plus tôt, la campagne a déjà eu lieu, les documents ont été distribués, tandis que l'on sait aujourd'hui tenir des bureaux de vote en respectant la distanciation sociale.

Si tel n'était pas le cas, le Gouvernement pourrait de nouveau solliciter le Parlement. L'avantage de notre proposition est qu'elle permet de borner le délai limite dans un temps plus court et de ne pas laisser les habitants de ces

Dans l'hypothèse, peu probable, où une vacance interviendrait aujourd'hui même, le délai maximum normal de trois mois conduirait à organiser des élections au plus tard le 8 mars, date à laquelle il est probable, selon le Président de la République, que nous ayons retrouvé nos restaurants préférés

a montré que les préfectures pouvaient s'adapter. Il ne nous paraît donc pas judicieux d'instaurer aujourd'hui un dispositif qui repousserait d'éventuelles élections sénatoriales partielles au-delà du mois de mars.

Trois éléments plaident en faveur d'un délai bref. D'abord, bon nombre de communes comptent moins de 1 000 habitants. Il ne s'agit donc pas d'espaces densément peuplés, et il est par conséquent plus facile d'y assurer le bon respect des gestes barrières, tant pour la campagne que pour le vote. Ensuite, il s'agit souvent de pourvoir au remplacement d'un ou de deux sièges vacants. De plus, dans les communes plus importantes, ces élections interviennent quelques mois après le renouvellement général et les forces en présence sont connues de la population. La campagne sera donc nécessairement différente et pourra s'adapter aux règles sanitaires.

Une date moins lointaine que celle prévue par le Gouvernement nous semble donc souhaitable. C'est pourquoi, comme pour les législatives partielles, nous proposons d'ajouter un délai supplémentaire de trois mois au délai de droit commun, soit six mois entre le fait générateur et la date ultime pour l'élection. Concrètement, si l'application du délai de droit commun de trois mois aboutissait à l'organisation d'une élection pendant l'état d'urgence sanitaire, le dispositif dérogatoire s'appliquerait. Au-delà du 16 février, le droit commun redeviendrait la règle. Il en irait de même pour les conseils d'arrondissement et les commissions syndicales. Pour finir, nous notons avec satisfaction que le Gouvernement a pris en compte les conséquences d'un allongement de la durée des campagnes électorales sur le plafonnement des comptes de campagne, en octroyant une majoration des plafonds de dépenses. La question des opérations de vote nous semble néanmoins imparfaitement traitée. Bien entendu, le principe de la double procuration est une bonne chose, et je salue également la proposition de Mme la rapporteure visant à permettre aux personnes vulnérables d'établir une procuration depuis leur domicile leur domicile sans justificatif. Néanmoins, je pense qu'il faudrait ajouter une expérimentation en matière de vote par correspondance ; c'est sans doute le moment.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la crise sanitaire inédite que nous devons affronter depuis le début de l'année a bouleversé notre vie sociale et durement éprouvé notre vie économique. Si elle a également des conséquences sur la vie démocratique de notre pays, elle a révélé la formidable capacité d'adaptation des élus, tant au niveau local qu'au niveau national, pour maintenir une écoute attentive des attentes de nos concitoyens. Toutefois, la circulation active du virus covid-19 sur l'ensemble du territoire et les risques importants de propagation de l'épidémie qui pourraient résulter de l'organisation de scrutins électoraux ont conduit à adapter, à plusieurs reprises, le calendrier électoral. Suivant l'avis du comité scientifique covid-19, mis en place auprès du Gouvernement, nous avons ainsi été amenés à reporter le second tour des élections municipales du 22 mars au 28 juin 2020, les élections consulaires de mai 2020 à mai 2021, et le renouvellement de six sénateurs représentant les Français de l'étranger pour permettre, au préalable, le renouvellement des conseillers et délégués consulaires qui composent leur collège électoral. L'élection de ces six sénateurs est ainsi reportée d'une année, soit à septembre 2021. Par ailleurs, aucune élection partielle pour les députés et les sénateurs des Français de l'étranger ne peut être organisée entre le 11 juillet et la date des élections consulaires de mai 2021. Aujourd'hui, la deuxième vague de l'épidémie commande des adaptations dans le fonctionnement de nos institutions nationales et locales. Cela a été le cas au Parlement, puisque les deux chambres se sont organisées pour siéger de manière continue, y compris au plus fort de la crise sanitaire. Cela a aussi été le cas dans les institutions locales- communes, intercommunalités, départements, régions -, qui ont mis en oeuvre les protocoles sanitaires et instauré différents modes de réunion afin de respecter au maximum les règles de distanciation physique et les gestes barrières. L'objectif impérieux était d'éviter la propagation du virus, tout en continuant de faire fonctionner les institutions. Dans ce contexte, les deux projets de loi, l'un organique, l'autre ordinaire, que nous examinons cet après-midi, prévoient la possibilité de reporter les élections partielles. Certaines d'entre elles sont déjà prévues, tandis que d'autres pourraient intervenir au cas où des scrutins, municipaux notamment, seraient invalidés. L'article unique du projet de loi organique prévoit la possibilité de reporter la tenue des élections partielles pour les députés et les sénateurs au-delà du délai de trois mois après la constatation de la vacance de leur siège, prévu par le droit en vigueur. L'organisation du scrutin interviendrait alors « dès que la situation sanitaire le permet », notamment au regard des recommandations du comité scientifique, et au plus tard le dimanche 13 juin 2021. Cet article s'appliquerait sur l'ensemble du territoire. Le projet de loi ordinaire prévoit, quant à lui, des dispositions semblables à son article 1 pour les élections partielles relatives à un siège de conseiller municipal ou de conseiller d'arrondissement et, à son article 2, pour les élections des membres des commissions syndicales. Deux dispositions introduites à l'Assemblée nationale sont à relever : un même mandataire pourra disposer de deux procurations, au lieu d'une seule comme le prévoit le droit en vigueur les plafonds de dépenses sont majorés de 5 % par mois pour tenir compte de l'allongement de la durée de campagne, si les conditions sanitaires ne permettent pas d'organiser l'élection partielle dans les délais de droit commun, à savoir trois mois pour l'ensemble des élections, à l'exception des élections partielles au sein des conseils d'arrondissement, pour lesquelles le délai est de deux mois. Ces dispositions, enrichies des amendements de notre commission des lois, doivent permettre de concilier au mieux les principes de sincérité du scrutin et de préservation de la santé publique. Pour toutes ces raisons, le groupe Les

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous voici réunis pour étudier l'inscription dans la loi de la possibilité de reporter des élections partielles, nouvelle conséquence de la crise sanitaire sur notre vie démocratique. Après le report du second tour des municipales au printemps dernier, puis le report de l'élection de six des douze sénateurs représentant les Français de l'étranger à la fin de l'été, notre pays est de nouveau en questionnement quant aux conditions de maintien des temps démocratiques à venir. L'incompréhension et l'incertitude suscitées par le délai entre les deux tours des municipales ont laissé des traces. Certes, les circonstances à l'époque n'ont peut-être pas permis d'anticiper suffisamment les risques que pouvait faire peser une telle épidémie sur l'exercice de la démocratie, mais la sincérité d'un scrutin à deux tours pouvait-elle être maintenue avec un si grand écart entre les deux Sans revenir sur les polémiques liées au choix du maintien des élections municipales- en tout cas du premier tour -lors de la première vague, la deuxième vague que nous vivons et l'évolution épidémiologique incertaine pour le premier trimestre 2021 nous obligent à intervenir afin de préserver à la fois le temps de la campagne et celui du vote. Les discussions que nous avons eues mettent bien en avant le motif impérieux d'intérêt général que constituerait le haut niveau de l'épidémie de la covid-19, qui devrait entraîner le décalage des élections prévues pour l'an prochain. Les deux textes que nous étudions en même temps sont donc guidés par un impératif lié à l'incertitude sanitaire des prochains mois, mais aussi par les règles interdisant l'organisation de scrutins législatifs au cours de l'année précédant l'expiration des mandats de député, à savoir le 21 juin 2022.

À ce jour, il n'y a que deux législatives partielles à organiser, mais l'élection d'une dizaine de nos collègues sénateurs fait toujours l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel, ce qui pourrait rendre nécessaire la tenue d'élections partielles.

Celles-ci nous sont certes plus familières, car pratiquées de longue date, mais elles restent néanmoins peu sûres et ne garantissent pas la sincérité du vote. Ce projet de loi nous est soumis alors que, d'ici peu, la traduction législative du rapport Debré sur la faisabilité des élections départementales et régionales sera sur le bureau du Sénat. ses conclusions, indique ceci : le scénario d'un report à la fin du mois de juin 2021, assorti d'une évaluation de la situation sanitaire- effectuée par le conseil scientifique et remise directement au Parlement avant la tenue des scrutins, est celui qui est susceptible de répondre au mieux aux contraintes sanitaires et de recueillir le plus large assentiment possible parmi les forces politiques du pays. Je souhaite attirer votre attention sur ce dernier point. Oui, la décision de convoquer les élections émane de l'exécutif, mais les discussions sur les textes actuels ont permis de mettre au jour l'importance pour les partis politiques d'être informés, en toute transparence et sans délai, sur d'éventuelles dates afin d'assurer la nécessaire préservation de l'équité entre candidats. La commission a, ce matin, fait le choix de se détacher de l'avis du conseil scientifique pour fixer la date des nouvelles élections. Elle a proposé de la déterminer en fonction des données chiffrées émanant des ARS. Afin d'avoir une vision plus territorialisée, ces rapports devraient être publics afin de permettre une bonne information de l'ensemble des acteurs des élections. Nous trouvons cependant qu'un certain flou persiste : qui analysera les critères bruts fournis par l'ARS pour évaluer la faisabilité sanitaire ? Quels critères seront retenus pour convoquer l'élection ?

Je crois que le Gouvernement a raison de venir devant le Parlement. Parfois, il cherche à l'éviter ; là, au contraire, il a ressenti le besoin de venir devant nous pour que nous traitions cette question très délicate du report des élections partielles et des modalités de ce report. À vrai dire, il n'est pas si facile de prendre une telle décision. Tout d'abord, il est exact que le Gouvernement- il l'a fait une première fois pour l'élection législative du Pas-de-Calais -peut invoquer la théorie des circonstances exceptionnelles pour reporter, malgré les termes impératifs de la loi, une élection partielle, y compris une élection législative. Toutefois, de nombreux scrutins sont en cause.

peut se dire que, dans une commune rurale d'un territoire qui ne serait que faiblement affecté par l'épidémie,

me semble sage, même si je souscris aux propositions qui ont été retenues par la commission des lois, sur la recommandation de notre collègue

la date des élections ne soit pas laissée à l'entière discrétion du Gouvernement ou de l'administration pendant une durée qui, à compter de ce mois de décembre, serait supérieure à six mois.

à la prévention des risques de propagation du virus. Si le scrutin peut être organisé dans de bonnes conditions sanitaires, alors il doit l'être.

Merci,